Je vous prie d'excuser l'absence du président du Sénat, retenu aux obsèques d'un ancien sénateur. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, tant celui des orateurs que celui du temps de parole. La parole est à M. Hervé Marseille, pour le groupe Union Centriste.

Dès avril dernier, mon groupe avait proposé d'annuler les charges des PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, cela afin de cibler la mesure sur les entreprises les plus affectées et de limiter son impact sur les finances publiques. On nous avait répondu à l'époque qu'un tel dispositif serait encore trop lourd pour le budget de l'État et de la sécurité sociale. Nous pouvons l'entendre. Pour autant, monsieur le Premier ministre, à l'occasion de l'un des derniers comités de contrôle et de liaison, j'avais déjà attiré votre attention sur ce sujet et vous m'aviez répondu que vous aviez ce dossier dans le viseur.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Marseille, je vous remercie de votre question qui me donne l'occasion de souligner après vous l'impact extrêmement fort

reconnu dans votre question -que le Gouvernement et le Parlement ont déployé des moyens d'accompagnement extrêmement massifs qui, en termes comparatifs, sont reconnus comme tels, au bénéfice

tant que la crise dure. Nous examinerons, notamment dans le cadre de la conférence du dialogue social que je réunirai la semaine prochaine, un certain nombre de ces dispositifs au regard de la situation économique et sociale. Vous m'avez interrogé plus particulièrement sur la question des dettes fiscales et sociales des entreprises. Permettez-moi de rappeler au Sénat que, sur le plan fiscal, ce sont près de 25 milliards d'euros qui n'ont pas été prélevés auprès des entreprises, qu'il s'agisse de reports ou de remboursements accélérés de créances,

le plan social, le soutien est historique puisque les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs les plus touchés ont bénéficié de mesures d'exonération qui ont donc acquis un caractère définitif. Ce sont ainsi près de 8 milliards d'euros de charges sociales qui

un fauteuil sur deux est libre. Ah ! Sous la haute autorité du président Larcher, nous respectons en ce lieu les normes sanitaires, et le Sénat n'est pas un foyer épidémique. Dans le respect des mêmes normes sanitaires, Dans le respect des mêmes normes sanitaires, soit la vacance d'un fauteuil sur deux, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous autoriser la réouverture des salles de cinéma, des salles de spectacle et des salles de concert ? En 2020, votre gouvernement a consacré près d'un milliard d'euros pour garantir les droits aux allocations des intermittents du spectacle. Cet argent aura été dépensé en pure perte si votre gouvernement ne met pas en place maintenant des aides spécifiques pour accompagner les artistes dans la reprise de leur activité. votre gouvernement, dans le cadre général d'une réforme de l'assurance chômage que nous dénonçons, a lancé une mission de réflexion sur le régime de l'intermittence et a souhaité notamment que soit étudiée sa convergence avec le régime général tel qu'il sera réformé pour pour « ne pas générer d'inégalités supplémentaires entre ceux-ci ». Le monde de la culture, avec d'autres, a été durement touché par la pandémie. Les artistes ont besoin d'un fort soutien de la Nation, d'être rassérénés par l'assurance de la pérennité d'un régime qui garantit leur existence. Monsieur le Premier ministre, la culture n'est pas accessoire, secondaire ou subalterne ; elle est essentielle, car elle constitue l'essence même de notre Nation.

l'occasion pour moi de rappeler quelques points de contexte. Premièrement- Olivier Véran y reviendra certainement en détail dans quelques instants -, la pandémie continue de toucher durement notre pays et l'Europe. Deuxièmement, les lieux culturels et les lieux de spectacle sont fermés pour 85 % des citoyens européens parce qu'on mène en Europe une politique de prévention.

solidarités et de la santé, nombre de nos concitoyens doivent renoncer à se soigner et sont ainsi privés de la possibilité de voir ou d'entendre correctement, parfois même de sourire. Ces difficultés d'accès aux soins entraînent chaque fois des drames individuels, comme le rappelait le Président de la République lors du 42 congrès de la Mutualité française. Lorsque les Français, faute de moyens, renoncent à une nouvelle paire de lunettes ou à un appareil auditif, c'est notre pacte social qui est abîmé. C'est pourquoi, dès 2019, le Gouvernement a mis en place la réforme du « 100 % santé ». Après les soins dentaires et l'optique l'an dernier, les aides auditives sont désormais prises en charge à 100 % depuis le 1 janvier 2021. Permettre aux Français, notamment les plus fragiles, d'accéder à des soins de qualité : telle est l'ambition de cette réforme de justice sociale. Nous en avons désormais la certitude : cette réforme porte ses fruits. Demain, jeudi 11 mars, paraîtra une étude Harris Interactive pour l'UFC-Que choisir et le réseau Santéclair montrant que 50 % des ventes d'appareils auditifs réalisées en janvier et en février de cette année ont porté sur des offres sans reste à charge. Cette réforme bénéficie à tous : aux Français, bien sûr, en premier lieu, mais aussi aux assureurs, aux mutuelles et aux professionnels, car tout en préservant la clientèle existante, un nouveau public accède désormais à des produits sans reste à charge. le Président de la République fait du en matière de santé une priorité absolue. Il s'agit de soutenir davantage nos PME françaises, mais également de faciliter les approvisionnements et de les rendre plus responsables. Il s'agit aussi de défendre notre souveraineté sanitaire, qui passera par un soutien à la production française de ces dispositifs médicaux qui sont désormais parfois le quotidien des Français. La création d'un label visant à mieux informer nos concitoyens et à les éclairer dans leurs choix constituerait à cet égard une piste de réflexion intéressante. Ma question est donc la suivante, le ministre Elle arrive ! Je sais que cela vous dérange ! Monsieur le ministre, comment rendre cette réforme plus lisible pour que les Français s'en saisissent pleinement tout en favorisant la production française et en soutenant nos PME ? Monsieur le ministre,

En 2021, dans la société française, les inégalités liées au travail sont bien réelles. L'écart salarial brut entre les hommes et les femmes est de 28 %. À l'heure de la retraite, les femmes perçoivent en moyenne une pension inférieure de 41 % à celle des hommes. Tel est le triste résultat des inégalités professionnelles et des carrières précarisées des femmes. Celui-ci s'explique par les temps partiels subis, par le fait que 80

87 % des aides-soignantes sont des femmes. Elles sont en première ligne pour prendre soin de nos aînés et des personnes vulnérables, puisque 97 % des aides à domicile sont des femmes. Elles sont majoritaires dans les métiers de l'éducation, de la grande distribution, dans le secteur de la propreté, métiers dits « essentiels Revalorisons ces métiers et nous ferons coup double : nous réduirons l'écart de rémunération et nous sortirons des préjugés et des stéréotypes existant sur ces métiers en tension qui intéressent aussi les hommes. Vous avez fait un premier pas avec le Ségur de la santé en revalorisant les carrières des professionnels de santé rattachés aux hôpitaux, mais vous en avez exclu, par exemple, les sages-femmes et tout le champ du social et du médico-social, dont les aides à domicile. les premières de corvée sont-elles les oubliées des premiers de cordée qui forment le cabinet présidentiel ? Êtes-vous prêt à revaloriser les métiers du social et du médico-social, qui représentent plus de 1 million de salariés, dont 175 000 postes à pourvoir à l'échelle nationale d'ici 2025 ? Donnez les moyens aux gestionnaires de ce secteur, quel que soit leur statut, de relever ce défi

en concertation avec les partenaires sociaux une revalorisation des métiers dits « de la deuxième ligne » : les hôtes et hôtesses de caisse, les éboueurs, les agents d'entretien, les aides à domicile, qui se sont tous mobilisés de manière exceptionnelle durant cette pandémie. Il faut conclure. En conclusion, madame la sénatrice, pour réaliser cette égalité économique pour réaliser cette égalité économique entre les femmes et les hommes, nous devons mener des politiques très volontaristes. Une proposition de loi a été déposée en ce sens à l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis. Le chemin vers l'égalité est encore long, ... Il faut vraiment conclure, madame

et de la santé, le message envoyé le dimanche 7 mars par la direction générale de la santé à propos de l'interruption des livraisons de vaccins pour une semaine aux généralistes au profit des officines a suscité la stupéfaction des médecins, de leurs patients, mais aussi des pharmaciens. Les personnes qui devaient être vaccinées la semaine prochaine dans les cabinets voient donc leur rendez-vous annulé, sans même savoir si les pharmaciens prendront le relais. À vouloir multiplier les vaccinateurs sans coordination, on ne multiplie ni les vaccins ni les vaccinés. Les enjeux définis sont la santé publique et son efficacité. Multiplier les acteurs et les centres de vaccination est évidemment un objectif louable. La vaccination s'est incontestablement accélérée, et c'est un point fort. Il est important de stabiliser l'organisation en place pour monter en puissance ensuite, car les professionnels et les citoyens ne comprennent plus ces changements de cap. Il y a un réel problème de méthode dans la gestion de cette crise sanitaire. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais de comprendre les décisions pour gagner en acceptabilité. Pourquoi ne pas passer par une organisation territoriale, comme vous l'avez fait pour les confinements avec l'appui des élus locaux, en permettant aux pharmaciens de vacciner, tout comme les infirmiers et les sages-femmes, dans les territoires dépourvus de médecins ou lorsqu'il n'y a pas assez de médecins volontaires, et non pas à leur place ? Cette décision va démobiliser les médecins engagés qui ont fait acte de citoyenneté en se mobilisant à vos côtés pour accélérer la vaccination. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer les motivations qui vous ont conduit à prendre cette décision ?

mesdames, messieurs les sénateurs, vous y serez sensibles, je remercie les médecins libéraux qui sont très nombreux à se mobiliser pour vacciner, mais la moitié d'entre eux n'a pas encore passé de commande. De ce fait, la moitié des Français ne peut toujours pas se faire vacciner dans son cabinet de ville. Nous avons donc considéré qu'en plus des médecins, il fallait permettre aux pharmaciens de commencer à vacciner pour permettre à tous les patients sur tout le

il faut arrêter d'infantiliser les Français. Sans explication des enjeux, ils ne peuvent pas comprendre les mesures. Comment comprendre qu'ils peuvent aller en Espagne ou en Italie et y manger au restaurant alors qu'en France, ces derniers sont fermés depuis six mois ? Comment comprendre qu'ils peuvent prendre le métro, le RER, le TGV et l'avion, mais qu'ils ne peuvent aller ni au cinéma ni au théâtre ?

dès 2014, la Chine accuse les Ouïghours, minorité musulmane du Xinjiang, de radicalisme politique et religieux et construit des camps dit « de rééducation » pour les y enfermer de manière préventive. Entre 1 et 3 millions d'Ouïghours sont déportés arbitrairement dans ces camps de concentration et de travail. Les enfants sont éloignés de leurs parents, les couples séparés. Les détenus doivent renoncer à leur langue et à leur religion. On y pratique stérilisations et avortements forcés. Les tortures et les viols sont le lot quotidien. L'objectif des autorités chinoises est d'éradiquer l'identité ouïghoure. Le 17 décembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution visant à sanctionner les responsables chinois à l'origine de ce nettoyage ethnique. Vous-même, monsieur le ministre, en février 2021, avez dénoncé « un système de répression institutionnalisé » devant le Conseil des droits de l'homme des Selon une étude australienne, des dizaines de milliers d'Ouïghours ont été transférés dans des usines appartenant à 83 grandes marques internationales, où ils sont en situation d'esclavage. Hier, au Conseil de Paris, le groupe écologiste déposait un voeu relatif à l'oppression des Ouïghours. du Sénat qui vous demande d'user avec d'autres membres de l'Union européenne de votre pouvoir de pression économico-diplomatique, si puissante que puisse sembler la Chine. Que comptez-vous faire ? Oserons-nous dire demain que nous ne savions pas ou que nous ne pouvions rien ?

vous avez évoqué avec justesse les pratiques injustifiables qui se déroulent au Xinjiang.

mon appel insistant pour qu'une mission impartiale, indépendante et transparente d'experts internationaux puisse se rendre dans le Xinjiang le plus vite possible, sous la responsabilité de la haute-commissaire aux droits de l'homme, Mme Bachelet. Je tiens aussi à rappeler la responsabilité des entreprises françaises, qui doivent exercer la plus grande vigilance possible, y compris en tant que sociétés mères, sur les risques liés à la chaîne de valeur et sur la nécessité de prévenir des atteintes graves aux droits fondamentaux des Ouïghours.

Partout dans nos campagnes, sur le bord des routes, nous voyons des poteaux abîmés et des lignes téléphoniques à même le sol. Les élus locaux sont démunis face à cette dégradation du réseau.

Monsieur le ministre, ma question concerne donc la maintenance de ce réseau. De nombreux élus locaux nous font part de situations déplorables, voire dangereuses, qui attestent le manque d'entretien du réseau en zone rurale. J'imagine que l'Ardèche n'y échappe pas. En Maine-et-Loire, dans Les Hauts d'Anjou, il a fallu la mobilisation des élus locaux pour que l'opérateur entretienne correctement le réseau. Monsieur le ministre, avez-vous dressé un état des lieux de la situation ? Quel suivi comptez-vous mettre en oeuvre pour garantir la maintenance du réseau cuivre jusqu'à sa disparition complète ?

le réseau cuivre doit s'éteindre en 2030 pour être remplacé par un réseau fibre. D'ici là, il est essentiel d'assurer son entretien. Nous avons tous et toutes pu constater, notamment dans les départements ruraux,

dont les réparations doivent être faites et dont le réseau doit être entretenu. Il posera les bases du futur service public universel intégrant le haut débit. Il fixera un calendrier et une carte de déploiement des travaux pour assurer l'entretien et l'accès à un réseau cuivre de qualité. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à travailler, tout particulièrement dans le cadre du plan de relance, sur le déploiement du très haut débit. Nous avons prévu des crédits supplémentaires à la fois pour les réseaux de fibre optique, mais aussi pour le déploiement de nouveaux pylônes, de façon à permettre un accès en tous lieux et dans de bonnes conditions à une solution de téléphonie. La parole est à M.

recul de la laïcité, mise en cause des professeurs, à Paris, à Grenoble et ailleurs. Le débat se focalise sur l'influence que peut avoir la convergence de l'islamisme radical et de l'extrême gauche, que certains qualifient d'« islamo-gauchisme », sur la vie quotidienne et les études dans dans les établissements d'enseignement supérieur. La simple utilisation de ce terme « islamo-gauchisme » pour décrire, même imparfaitement, un phénomène réel vous expose déjà, madame la ministre, à des procès en sorcellerie. Vous avez pris le parti- et c'est courageux -de vous saisir du problème, et vous avez commandé un bilan de la recherche, demande aussitôt qualifiée par des chercheurs et syndicats de « menace de répression intellectuelle Je note qu'une partie de l'exécutif a pris ses distances avec votre initiative, évoquant « l'attachement absolu du président de la République à l'indépendance des enseignants-chercheurs ». Ma question est simple : peut-on faire du « en même temps » sur ces sujets graves ? Quelle est la véritable doctrine du Gouvernement en la matière ? D'ailleurs, y en a-t-il une ? La parole est à Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

quelle quantité d'universitaires empêchés, quelle réelle pluralité sur les sujets de recherche ? C'est en affrontant ces questions que nous préserverons la liberté académique de tous, ce qui est essentiel Pascal Allizard, pour la réplique. L'enseignement- je le crois, et je pense que nous en sommes tous convaincus -est, et doit rester, le creuset de la République et de la Nation. On ne peut pas accepter sans réagir qu'il devienne l'incubateur du séparatisme, non plus que de voir des enseignants placés sous protection policière. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est aussi cantonner la religion, quelle qu'elle soit, à la sphère privée,

La semaine dernière, mon collègue Jean-François Husson interrogeait le Gouvernement sur les délais de remboursement partiel des masques achetés par les collectivités. Force est de constater que, dans mon département, 25 % des communes sont toujours en attente. Je souhaite nous donner l'occasion, cet après-midi, d'anticiper sur le remboursement des charges liées aux centres de vaccination.

: « Cela fonctionne bien ! » Cela fonctionne bien grâce à la mobilisation de tous, qu'il s'agisse des agences régionales de santé, des préfets, des élus, des agents des collectivités territoriales, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des sages-femmes, des retraités ou des étudiants. Il faut le dire. tous la formule consacrée du « quoi qu'il en coûte ». Elle s'applique aussi au fonctionnement des centres. Nous adapterons le soutien financier aux municipalités, de manière à les accompagner dans la durée, et encore plus dans la phase d'accélération de la vaccination.

pourront ainsi financer les dépenses les plus urgentes des 1 300 centres ouverts sur le territoire national. Nous travaillons à l'élargissement et à l'assouplissement du financement que nous apportons aux structures qui ne sont pas encore labellisées. Ces 60 millions d'euros ne correspondent pas à un solde de tout compte, madame la sénatrice, mais ils sont une amorce importante. Ils seront réabondés autant que nécessaire. Le financement des centres n'est pas, ne sera pas et ne devra pas être, à aucun moment, un facteur bloquant dans la campagne de vaccination, à laquelle tout le monde oeuvre avec beaucoup de courage sur tout le territoire national. La parole

pour les différents postes

sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques, particulièrement dans le domaine des transports. En 2018 et 2019, le Conseil constitutionnel a censuré par deux fois vos chartes facultatives, sur l'initiative du groupe parlementaire socialiste. Le 4 mars 2020, la Cour de cassation a requalifié un chauffeur Uber en salarié, qualifiant sa situation d'« indépendance fictive » ! Le 30 novembre 2020, le rapport Frouin, que vous avez commandé, a enterré l'idée d'un tiers statut.

afin que la justice vous contraigne à solliciter l'inspection du travail. Mais où est donc passé l'État de droit ? Madame la ministre, allez-vous enfin saisir l'inspection du travail pour protéger ces travailleurs plutôt que les plateformes ?

C'est la raison pour laquelle la ministre du travail, que vous avez citée à de nombreuses reprises, a nommé trois personnes qualifiées pour mener des concertations avec ces acteurs.

ailleurs, la ministre du travail réunira les partenaires sociaux, vendredi prochain, pour aborder ce sujet dans le cadre du groupe de travail paritaire de l'agenda social sur les formes particulières d'emploi.

des solidarités et de la santé, après l'année terrible que nous avons vécue, l'arrivée de vaccins contre le virus laisse entrevoir un espoir, celui d'un retour à la vie normale que les Français, malgré leur discipline, leur solidarité et leur remarquable patience, n'en peuvent plus d'attendre. Tous nos soignants se sont mobilisés pour protéger la population, et parmi elle les personnes les plus fragiles. Pour ma part, j'ai oeuvré dans un centre de vaccination pour personnes handicapées, le week-end dernier ; et je me suis réjouie de constater, comme partout ailleurs sur le territoire, une nette augmentation des capacités de vaccination. Je crains néanmoins, à la lumière de ce qui a suivi, que les événements de ce week-end ne soient qu'une accélération en trompe-l'oeil. L'implication générale de tous les acteurs tranche avec l'image que renvoient la DGS et son directeur, qui n'a cessé d'enchaîner les imprécisions et les décisions contestables et contestées.

L'un de nos collègues, médecin de profession, peut témoigner de l'annulation de 200 rendez-vous ! Il s'agit, au mieux, d'un couac qui ne sera pas le premier dans la gestion de cette épidémie. À chaque jour sa nouvelle stratégie : c'est insupportable Monsieur le ministre, nous n'avons tous qu'un seul souhait : celui que la campagne de vaccination s'accélère. Nous disposons d'une force de frappe considérable qui ne demande qu'à être sollicitée, au premier rang de laquelle les médecins, mais aussi les pharmaciens et les pompiers, dont la mobilisation pourrait permettre de multiplier par dix les capacités de vaccination. Aussi, je vous le demande, monsieur le ministre : pourquoi avoir laissé la DGS infliger un tel camouflet aux médecins généralistes, si ce n'est pour masquer une nouvelle pénurie ?

commandés par des médecins libéraux en vue d'être injectés à leurs malades pour les protéger. Si je fais le calcul avec vous, sur ces 1,6 million de vaccins qui auront été reçus à date de vendredi soir, environ 450 000 auront été injectés, de sorte

Comme vous le savez, monsieur le ministre, la Nouvelle-Calédonie est actuellement en proie à une série de crises. Crise institutionnelle et politique, après le renversement du gouvernement il y a un mois. L'actuel gouvernement ne parvient pas à se trouver un président, à la veille d'une probable demande de troisième référendum sur l'indépendance. Crise budgétaire, puisque le territoire doit voter son budget avant le 31 mars, sous peine d'être placé sous tutelle de l'État. Crise industrielle et économique, avec un cours du nickel à son étiage et le conflit relatif à la vente de l'usine du Sud, qui heureusement semble aujourd'hui résolu. catastrophe naturelle liée au passage du cyclone Niran. Enfin, la crise est aussi sanitaire, avec la détection des premiers cas de covid dans ce territoire qui jouissait jusque-là de son statut privilégié de zone, et qui se retrouve entièrement confiné depuis lundi. L'impression générale qui se dégage est alarmante. Ce sont les dix plaies d'Égypte ! Monsieur le ministre, la France n'est pas seulement l'Hexagone ; c'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Face à cette situation exceptionnelle, les réponses de l'État sont-elles à la hauteur ? Avez-vous pris la mesure de la crise que traverse le territoire néo-calédonien ? Quelle est votre stratégie pour y remédier ? La parole

le Gouvernement est bien sûr prêt à discuter, y compris d'un nouvel accord, puisque nous savons très bien qu'il faut désormais écrire les lendemains de l'accord de Nouméa. Voilà, en quelques mots et en deux minutes, ma réponse aux dix plaies d'Égypte que vous avez évoquées pour la Nouvelle-Calédonie, pour le Caillou.

Si les affrontements entre groupes de jeunes existent depuis longtemps, nous sommes en train d'assister à une explosion inédite de la délinquance de rue et de la violence juvénile. Rien que cette semaine, plusieurs jeunes de moins de 15 ans ont été grièvement blessés. Et c'est tous les jours que l'on assiste à un événement dramatique ! Cette nuit encore, à la veille de cette séance de questions d'actualité au Gouvernement, en plein coeur du XVI arrondissement de Paris, dans un quartier pourtant réputé calme, des affrontements violents Il est hors de question de s'abandonner à la fatalité ni de laisser s'installer une sorte de résignation collective. Laisser croire que l'on a tout essayé n'est pas acceptable Monsieur le ministre, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à rétablir l'ordre. Les policiers sont épuisés et héroïques, mais on a le sentiment qu'il est plus facile pour la préfecture de police d'évacuer les berges de la Seine que de lutter contre la délinquance de rue. Très bien ! Le 27 janvier que la tension montait, notamment à la porte de Saint-Cloud, où j'ai assisté à des heurts. Un mois et demi après, toujours pas de réponse ! Lorsque vous le croiserez, monsieur le ministre, n'hésitez pas à lui remettre ce courrier, que je tiens à votre disposition.

Ma question est simple : quelles mesures opérationnelles comptez-vous mettre en oeuvre immédiatement pour que les villes ne deviennent pas le terrain d'affrontements systématiques de jeunes armés jusqu'aux dents, sur fond de revendication de territoires et de réseaux sociaux ? La parole

Je suis d'accord pour travailler avec vous, mais ne confondons pas les violences urbaines sur fond de règlements de comptes et ce qui peut se passer, et qui est effectivement tout à fait déplorable, pour des enfants de 11 ou de 12 ans.

En effet, la grande majorité des 225 millions de doses de vaccins ont été administrées dans quelques pays riches et producteurs de vaccins, tandis que la plupart des pays à revenus faibles ou intermédiaires attendent encore. l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et relayé par le Président de la République Emmanuel Macron, les pays du G7 se soient engagés à partager une partie de leurs vaccins et à verser des sommes importantes pour financer le mécanisme Covax. Sur ce point, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer précisément quel est le décaissement réel effectué par la France sur sa contribution financière aux différents programmes de vaccins destinés aux pays du Sud ?

Aussi, monsieur le ministre, afin de mettre ses actes en conformité avec ses déclarations et d'amplifier l'ambition du mécanisme Covax, le gouvernement français est-il prêt à soutenir l'initiative indo-sud-africaine pour une levée des barrières protégeant les brevets des vaccins anti-covid-19 ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Gilbert Roger, vous avez raison, la solidarité internationale

les maisons d'arrêt sur le plan national. Vous vous en êtes vous-même inquiété. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le nombre de détenus a connu une chute historique, qui n'est malheureusement pas liée à une baisse de la délinquance, mais au double effet du quasi-arrêt des juridictions pendant le confinement et des mesures de libération exceptionnelles prises pour

150 % à Villepinte. Comment s'étonner, dès lors, que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France en utilisant les mots « dégradant » et « inhumain » ? Monsieur le ministre, cette situation n'honore pas notre pays. Nous avons bien compris que votre souhait est d'instaurer un carcéral et que, pour vous, malgré l'augmentation de la délinquance, c'est le quantum des peines qui devra s'adapter au nombre de places de prison. Le Président de la République avait promis la création de 15 000 places de prison pendant son quinquennat. Si les objectifs annoncés avaient été tenus, on ne parlerait peut-être pas de surpopulation

Il en est ainsi décidé. Par lettre en date du 5 mars 2021, M. Patrick Kanner, président du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, demande l'inscription à l'ordre du jour d'un débat sous la forme d'une série de questions-réponses

l'examen de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels étant de ce fait reporté à l'issue de ce débat. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. En conséquence, nous pourrions avancer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance sur cette proposition de loi, initialement prévu à l'ouverture de la discussion générale, au même jour à quatorze heures trente. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux avant toute chose saluer cette initiative portée avec courage et détermination

un fervent défenseur de la décentralisation et des libertés locales. Je n'ai nul besoin de vous le rappeler ici : la compétence en matière d'eau et d'assainissement relève depuis la fin du XIXsiècle du bloc communal, responsable du bon fonctionnement de ce service. Pourquoi le législateur

Je sais que cela ne plaira peut-être pas à certains, mais je le rappelle : l'État n'est pas compétent. Toutefois, il est présent et prend sa part, tant dans les réparations d'urgence- près de 6 millions d'euros ont été mobilisés rien que l'année dernière pour résorber plus de 4 000 fuites

adéquate. Ce texte n'a pas pour objet de priver les élus locaux de leurs prérogatives, mais bien de construire les bases saines d'une nouvelle gouvernance de l'eau dans un milieu insulaire et de poser la première brique pour offrir à nos concitoyens un service de qualité, sans oublier les attentes en la matière sur le plan écologique. pour objet de suivre le chemin tracé par les élus locaux, notamment ceux des EPCI, qui s'accordent depuis plus de cinq ans sur le principe de la création d'une structure unique. Ils me l'ont d'ailleurs tous confirmé lors de nos échanges, que ce soit par courrier, en visioconférence ou lors de mon déplacement en Guadeloupe à la fin de l'année dernière. La commission départementale de la coopération intercommunale de la Guadeloupe, qui s'est réunie le 4 mars dernier, a une nouvelle fois témoigné de cette volonté des élus, mais certains sujets ne font toujours pas consensus. Je veux ici être clair et transparent : les deux initiatives, l'initiative parlementaire que nous discutons ici et l'initiative locale, ne sont ni en concurrence ni en contradiction. Jamais la question de la gouvernance de l'eau en Guadeloupe n'a autant avancé que depuis ces derniers mois.

Pendant plusieurs années, la gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe n'a pas été à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Environ 100 000 usagers sont régulièrement victimes de « tours d'eau ». Les syndicats compétents sont pour la plupart dans des situations difficiles, qui ne leur permettent ni d'effectuer les travaux d'urgence, ni de faire les investissements nécessaires à l'amélioration et l'entretien du réseau, ni de payer leurs fournisseurs. Cette structure unique aurait pour objet de répondre à ces défaillances en mettant tout le monde autour de la même table, au nom de l'intérêt général. Cette démarche est synonyme de mutualisation des capacités d'investissement et de fin des conflits autour de la gestion des ressources. La proposition de loi prévoit donc de créer le syndicat unique que nous appelons tous de nos voeux, élus locaux, parlementaires et Gouvernement. Je le répète, cette structure est une condition nécessaire, mais elle n'est qu'une première étape. Les collectivités devront pleinement s'emparer de ce nouvel outil, pour qu'il puisse réellement répondre aux attentes des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Que les choses soient claires : les élus locaux restent compétents en la matière.

Autre évolution, les usagers trouvent toute leur place dans ce nouveau schéma de gouvernance avec la création d'une commission de surveillance. Nous le savons, il s'agissait d'une demande forte des usagers de l'eau : être davantage associés à cette gouvernance. Je crois en la démocratie représentative. En ce sens, celui qui décide est responsable. Il est donc élu. La loi Engagement et proximité, que j'ai défendue ici même en 2019, a d'ailleurs eu l'occasion de réaffirmer ce principe, en réservant par exemple aux seuls élus la possibilité de participer aux délibérations des comités syndicaux. Ainsi, les parlementaires ont prévu de créer une commission de surveillance, qui rassemblera la société civile- les chambres consulaires, les représentants d'associations de protection de l'environnement -, les élus locaux- votre rapporteur y a veillé -et, bien sûr, les usagers, qui devront être majoritaires. Ce schéma, Ce schéma, précisé et renforcé par les deux assemblées, permettra d'associer durablement ces derniers dans la gouvernance. Il prévoit une commission de surveillance aux pouvoirs étendus, tout en conservant leur indépendance. Le président de la commission de surveillance pourra également participer aux travaux du comité syndical, avec voix délibérative. La création du syndicat mixte unique est évidemment une étape nécessaire. Je sais que des interrogations persistent sur la mise en place de ce syndicat, notamment à propos des personnels ou encore des dettes. Une préfiguration de l'organisation du nouveau service doit être expérimentée à l'échelon local. Les premières réflexions sur le modèle de ce syndicat unique ont été conduites dès 2018, avec un accompagnement financier de l'État. La préfiguration doit poursuivre ses travaux ; l'État est prêt à l'accompagner financièrement et à s'impliquer dans la réflexion. J'ai d'ailleurs eu de premiers échanges sur ce sujet- ils étaient épistolaires, pour la plupart -avec le président du conseil régional, Ary Chalus, et la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin. Selon moi, il existe plusieurs préalables à cette préfiguration, et ce afin d'avancer dans les meilleures conditions possible. La préfiguration doit être portée par une structure jugée légitime par tous au niveau de l'ensemble du périmètre concerné.

avec un regard neuf. Nous ne pouvons pas repartir comme avant, au risque que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour être très clair, car je sais que cela a peut-être été mal compris, cela signifie-t-il que les cadres actuels doivent être exclus des travaux ? La réponse est naturellement non. Cela signifie-t-il que les coordinateurs doivent nécessairement être issus de l'extérieur, c'est-à-dire ne pas être issus de la Guadeloupe ? Évidemment non. La Guadeloupe dispose d'une expertise locale, de compétences et de talents qui ont tout leur rôle à jouer dans ce combat sociétal qu'est devenu l'accès à l'eau. Et je ne doute pas que les usagers de l'eau en seront satisfaits. La préfiguration doit enfin associer l'État, qui pourra notamment mettre en oeuvre ses compétences dans plusieurs domaines. En parallèle, il est évidemment nécessaire d'anticiper la question de la prise en charge des dettes auprès des À l'Assemblée nationale, vos collègues députés ont adopté un amendement du Gouvernement tendant à transférer à la nouvelle structure unique les dettes bancaires, et uniquement celles-ci, afin de ne pas compromettre la viabilité de la nouvelle structure.

Je me suis engagé, et je m'y engage de nouveau, à ce que cette dette demeure soutenable pour les EPCI qui auront évidemment un rôle primordial dans la nouvelle structure. Deux solutions

ou les lycées, qui ont provisionné les fonds, mais aussi d'accompagner les nombreux usagers privés, qui souhaitent payer leur facture pour se mettre en règle et être tranquille d'esprit, mais qui en contestent le montant. L'État s'est d'ailleurs engagé à financer la pose de nouveaux compteurs d'eau dans l'un des EPCI, à sa demande.

La seconde solution consiste à développer des solutions innovantes, au cas par cas, pour les EPCI qui le souhaitent, avec les financeurs publics, l'AFD et la CDC, qu'il s'agisse d'un moratoire sur des prêts bancaires ou encore de la transformation de la dette due aux fournisseurs en dette bancaire.

À l'issue du dialogue social conduit avec les EPCI et le Siaeag, les personnels des services de l'eau actuellement en poste ont vocation, soit à être repris par le syndicat unique, soit à rester dans les EPCI, soit à partir pour ceux qui sont volontaires au départ, notamment à la retraite. Un état des lieux approfondi des ressources humaines a été conduit en 2019 et 2020. En ce qui concerne le Siaeag, soit 138 agents, un audit spécifique a été financé par l'État pour faciliter le reclassement des agents ou l'accompagnement des agents volontaires au départ. Par ailleurs, des entretiens des entretiens et ateliers ont été menés avec les équipes du Siaeag, des EPCI et les organisations syndicales en janvier 2021. Il est également important que le nouveau syndicat dispose d'une masse salariale en adéquation avec ses besoins, afin notamment de ne pas peser trop fortement sur la facture d'eau payée par les usagers. Vous le voyez, avec cette proposition de loi et les initiatives locales, nous tous, État, parlementaires, élus locaux, usagers, faisons un pas vers l'avenir. Un long travail reste à faire sur le terrain. Je sais pouvoir compter sur toutes les bonnes volontés, au Parlement ou au niveau local, pour nous rassembler autour d'un objectif commun auquel les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens aspirent avec force,

Face à un problème d'une telle gravité, l'action des pouvoirs publics est impérieuse : nous ne pouvons pas tolérer que nos compatriotes soient soumis à une telle indignité. Dommageable pour le tissu économique local, source de difficultés majeures de fonctionnement

De ces difficultés de gestion me semblent découler l'ensemble des difficultés que connaissent les Guadeloupéens dans leur accès à une eau potable de qualité. Ainsi, le réseau, qui court sur le territoire de plusieurs autorités gestionnaires, est mal connu, mal entretenu et partant de piètre qualité. En résultent des pertes massives. La gestion financière, qu'il est difficile de qualifier autrement que de catastrophique, obère toute capacité d'investissement et de remise en état de ce réseau. Enfin, la multiplicité des modes de gestion et des autorités gestionnaires empêche ces dernières de bénéficier d'économies d'échelle permises par la mutualisation des coûts. La solution à ce problème aux multiples causes est donc connue de longue date : il est impératif d'unifier la gouvernance de la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Les auditions que j'ai conduites m'ont d'ailleurs permis de constater le large consensus qui s'est construit autour du principe de cette unification en matière de gouvernance. Je comprends que les modalités pratiques de cette opération constituent, depuis plusieurs années, un point d'achoppement. l'esprit de solidarité et de consensus doit prévaloir sur ce sujet, dont la gravité nous oblige. Cette proposition de loi traduit une volonté d'apaisement, de concertation et de confiance dans l'intelligence du terrain : c'est d'ailleurs dans cette dynamique que j'ai souhaité inscrire mes travaux. Le présent texte me semble ainsi apporter une solution pragmatique à ce problème persistant. Par son article 1, il crée un syndicat mixte dit « ouvert », associant la région de Guadeloupe, le département de la Guadeloupe et les cinq communautés d'agglomération que compte la Guadeloupe continentale. Doté de missions étendues et cohérentes, ce syndicat mixte verrait le jour le 1 septembre 2021. Cette échéance m'a paru constituer un point d'équilibre satisfaisant entre l'exigence de célérité pour une structure trop longtemps attendue et le temps nécessaire aux préparatifs de préfiguration du syndicat mixte. Les statuts du syndicat mixte seraient arrêtés par le préfet de la Guadeloupe, après avis des organes délibérants des futurs Je sais la méfiance que peut susciter une telle procédure. Elle me semble nécessaire, cependant, en ce qu'elle manifeste la nécessité d'une impulsion de l'État sur ce sujet épineux. elle ne doit pas se traduire par un défaut d'association des élus locaux, et je sais combien notre assemblée sera, à juste titre, vigilante sur ce point. Lors de son examen en commission des lois, l'article 1 de cette proposition de loi a par ailleurs fait l'objet d'assouplissements qui me semblent bienvenus : la création d'une procédure d'adhésion au syndicat mixte, conditionnée à l'autorisation expresse du préfet de département et à l'accord unanime des membres préexistants, me semble opportune afin que nous ne soyons pas contraints, à l'avenir, de modifier la loi pour entériner un consensus local. De même, la possibilité pour le comité syndical de décider, à l'unanimité de ses membres, de déroger à la répartition des contributions financières me paraît de nature à faciliter et à fluidifier le fonctionnement de la future structure. La principale originalité de cette proposition de loi réside dans la création, par son article 2, d'une commission de surveillance ayant pour mission de formuler des avis et propositions sur l'activité du syndicat mixte nouvellement créé. Je sais la profonde défiance des Guadeloupéens envers leurs services publics d'eau et d'assainissement : les auditions que j'ai menées m'ont permis de constater le vif mécontentement qu'expriment les usagers de ces services. Trop Trop longtemps tenus à l'écart d'une situation qui affecte pourtant leur quotidien, ils doivent être associés, autant que faire se peut, au fonctionnement du nouveau syndicat mixte. La composition de la commission de surveillance garantit à leurs représentants, non seulement permettra, je le crois, une juste représentation de leurs intérêts et leur pleine association aux décisions du syndicat mixte. L'examen de cet article en commission a été l'occasion de parfaire la composition et le fonctionnement de ladite commission de surveillance. Ainsi, la présence des parlementaires guadeloupéens en son sein ne me semblait pas nécessaire. Nos collègues guadeloupéens, Victoire Jasmin, Victorin Lurel et Dominique Théophile, étaient d'ailleurs du même avis. Nous avons préféré assurer une meilleure représentation des élus municipaux. Par ailleurs, nous nous sommes Par ailleurs, nous nous sommes attachés à renforcer les prérogatives du président de cette commission de surveillance, qui, je l'ai dit, sera un représentant d'usagers. L'équilibre trouvé entre la représentation adéquate des intérêts des usagers et le fonctionnement fluide de la nouvelle structure me semble dès lors satisfaisant.

tant les questions qui resteront à régler sont nombreuses. Je déplore en particulier l'inertie de l'État sur ce sujet. Monsieur le ministre, je sais bien que l'État n'est pas resté passif : il a multiplié les interventions ponctuelles pour répondre à des situations de crise. Pourtant, comment se satisfaire de cette succession d'initiatives quand le problème structurel de la gestion défaillante des services était connu de tous, et de si longue date ?

À cet égard, cette proposition de loi n'a pas vocation à résoudre définitivement des questions comme le transfert au syndicat mixte des dettes, des ressources humaines et des biens nécessaires à l'exercice de ses compétences. Ce chantier exigera un dialogue particulièrement nourri entre l'ensemble des parties prenantes. ces questions auraient gagné à être résolues en amont, ce qui aurait grandement favorisé l'acceptabilité de la création du syndicat mixte unique. Monsieur le ministre, l'État doit donc se montrer à la hauteur de l'enjeu et jouer pleinement le rôle de facilitateur qui lui incombe. Vous pouvez compter sur notre vigilance.

Mme Justine Benin, rapporteure du texte à l'Assemblée nationale, et M. Dominique Théophile pour la qualité du travail accompli en commun, en Guadeloupe comme à Paris, pour sensibiliser sur la gravité de ce sujet et formuler des pistes de solution. Je ne doute pas que ces pistes recueilleront, à travers l'adoption de cette proposition de loi, une large adhésion, au Sénat comme à l'Assemblée nationale ! La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cette après-midi concourt à répondre à un problème crucial : celui de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. L'île se trouve en effet confrontée à des coupures d'eau fréquentes et à de multiples incidents sur le réseau. Parfois aléatoires, ces coupures sont aussi organisées sur certaines parties du territoire sous la forme de « tours d'eau » suscitant colère et exaspération. Les prestations servies aux usagers guadeloupéens ont de multiples conséquences sociales, économiques et environnementales. Cette situation est d'autant plus difficile à accepter qu'elle ne résulte pas de causes naturelles propres à la Guadeloupe, où la ressource en eau est abondante- M. le ministre L'un des principaux problèmes réside dans le caractère éclaté de la gestion des services d'eau et d'assainissement, qui fait obstacle à la gouvernance d'ensemble dont la Guadeloupe a impérieusement besoin. L'article 1 de la proposition de loi prévoit la création, au 1 septembre 2021, d'un établissement public régi pour l'essentiel par les dispositions applicables aux syndicats mixtes ouverts. Ses membres comprendraient, outre les cinq communautés d'agglomération de Guadeloupe continentale, le conseil départemental et le conseil régional. Les statuts du syndicat mixte ouvert seraient établis par le préfet, après avis des organes délibérants des collectivités territoriales et groupements concernés. serait dotée d'un bloc de compétences cohérent, axé sur la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées, du service de défense extérieure contre l'incendie et des eaux pluviales urbaines. Elle serait administrée par un comité syndical doté de vingt-huit délégués, soit quatre par membre. L'article 2 de ce texte prévoit la constitution d'une commission de surveillance auprès du syndicat mixte, chargée de l'organisation des procédures de transparence et d'association des usagers aux mesures prises par le service public de l'eau en Guadeloupe. La commission des lois a renforcé la solidité juridique du dispositif, en apportant des simplifications et améliorations rédactionnelles au texte. Nous pouvons nous en féliciter. Je me réjouis également de l'apport, par la commission des lois, d'un certain nombre d'assouplissements. Ainsi, alors que l'article 1 instaure une répartition rigide des contributions financières aux investissements consentis par le syndicat mixte ouvert, la commission a-t-elle prévu la possibilité pour les membres de décider, à l'unanimité, de déroger à la clé de répartition de ces contributions.

membres. Elle s'est également attachée à fluidifier le fonctionnement de la commission de surveillance. Elle a par ailleurs jugé utile de compléter les obligations du comité syndical à l'égard de la commission de surveillance, à celle-ci une audition annuelle du président du comité syndical. Enfin, elle a souhaité renforcer le rôle du président de la commission de surveillance en prévoyant qu'il pourrait, sur sa seule initiative, solliciter l'inscription d'une question à l'ordre du jour du comité syndical et qu'il disposerait d'un pouvoir de proposition d'audition à la commission de surveillance. Monsieur le ministre, chers collègues, cette proposition de loi constitue un premier pas vers la résolution d'une situation complexe et inacceptable pour les Guadeloupéens. Il paraît primordial d'élaborer rapidement une réponse concrète et pragmatique. Les élus du groupe Les Indépendants

mes chers collègues, la situation de l'eau en Guadeloupe est un problème à bien des égards : citoyens sujets à de nombreuses coupures d'approvisionnement, dépenses trop importantes, gaspillage de la ressource en eau, non-entretien du réseau, dette abyssale des structures gestionnaires, tarification et facturation opaques, Le constat de carence du système actuel est dressé par les acteurs institutionnels locaux et par l'ensemble des habitants, même si l'ambition de résilience climatique qu'il devrait appeler l'est peut-être moins.

En 2016 le volume d'eau consommée était de 26,4 millions de mètres cubes, alors que 73,1 millions de mètres cubes étaient produits. » Les pertes représentent donc 177 % de la consommation en eau de ces experts sont sans appel : pour un litre d'eau consommé en Guadeloupe, un litre et demi d'eau est perdu, ce qui entraîne bien entendu un stress trop important sur les ressources comme les eaux souterraines du Nord Grande-Terre. Surtout, la qualité de l'eau est « inquiétante », en raison

L'article 1 prévoit la mise en place d'une seule autorité, sous une forme proche d'un syndicat mixte dirigé par un comité syndical. Reste à espérer que cette unification soit soutenue par l'ensemble des acteurs politiques locaux : la représentation des différentes communautés d'agglomération ou des conseils départementaux et régionaux va dans ce sens. Toutefois, nous proposerons un amendement visant à permettre la présence de personnes qualifiées et de représentants d'usagers au sein même du comité syndical. Les graves problèmes qu'a subis la population appellent une implication forte des représentants des usagers au sein de cette nouvelle entité. doivent pouvoir, au même titre que des personnes qualifiées, non seulement observer, mais participer pleinement aux décisions prises par la nouvelle institution. Je note aussi que l'article 1 prévoit le transfert des dettes actuelles des organismes défaillants au nouveau syndicat mixte.

L'article 2 prévoit quant à lui la constitution d'une commission de surveillance, dans un souci de dialogue et de transparence avec l'ensemble des acteurs concernés. J'y insiste : selon nous, ce progrès n'est pas suffisant, mais il mérite d'être salué. Si la commission a permis des apports, notamment le renforcement des obligations du comité syndical, avec l'audition obligatoire annuelle de son président, nous souhaitons que cette instance puisse

à la forme que doit prendre cette nouvelle gouvernance et aux modalités de transition entre les deux systèmes, je reste à la fois enthousiaste et prudent. Oui, cette réforme est plus que nécessaire, et elle est vivement attendue. Oui, l'enjeu de l'eau doit être au coeur des réflexions de nos politiques publiques en général. Mais ce vaste travail nécessitera un engagement financier fort de l'État.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons cette après-midi rénove la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. La situation, vous la connaissez : ce sont des fuites à répétition et un réseau de distribution vétuste, qui demande d'importants travaux de renouvellement ; ce sont des coupures et des « tours d'eau » qui lassent, voire exaspèrent, alors même que cette ressource est abondante dans Pour ne citer que quelques chiffres, rappelons que le potentiel d'eau disponible par habitant y est d'en moyenne 7 000 mètres cubes, contre 3 000 dans les départements européens. Pourtant, l'eau ne coule pas toujours : la faute en revient à un réseau dont le rendement est largement inférieur à 50 %. Des pans entiers de l'économie s'en trouvent fragilisés,

Cette revendication, c'est la création d'une structure unique consacrée à la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, qui réunisse l'ensemble des communautés d'agglomération de Guadeloupe continentale, le département et la région. Cette structure, qui prendra la forme d'un syndicat mixte ouvert, est évidemment un préalable à la remise en état du système de distribution d'eau potable en Guadeloupe. Elle permettra d'en finir avec une organisation devenue progressivement trop complexe pour être efficace et trop atomisée pour apporter une réponse à la crise. C'est aussi la condition pour sortir- enfin ! -de l'impasse dans laquelle les erreurs et les manquements du passé nous ont conduits. Mes chers collègues, le texte qui vous est proposé aujourd'hui est le fruit d'un travail de longue haleine. Il prend ses racines dans la mobilisation des citoyens et des élus qui ont saisi ce sujet à bras-le-corps. Il a trouvé sa forme au cours de l'audition des élus, des représentants d'associations et de collectifs d'usagers, ainsi que des nombreux acteurs impliqués dans ce dossier. À l'Assemblée nationale, divers amendements ont permis d'améliorer et de préciser son dispositif. La création d'une commission de surveillance, en lieu et place de la commission consultative envisagée, garantira par exemple la juste représentation des usagers et permettra de restaurer une confiance perdue.

souhaité dépassionner ce débat. Nous avons voulu l'aborder avec une hauteur de vue qui privilégie la technicité et le dialogue, en nous débarrassant des contingences politiciennes qui ont trop souvent fait obstacle. Nous saluons tous ceux qui ont compris et favorisé cette démarche. Nous tenons également à saluer l'engagement du ministre des outre-mer dans ce dossier et sa volonté sans cesse renouvelée d'aller vite, qui est aussi la nôtre. « Là où il y a une volonté, il y a un chemin

à adopter en l'état cette proposition de loi, pour offrir enfin aux Guadeloupéens des services publics d'eau potable et d'assainissement à la hauteur de leurs attentes ! La parole

la gestion du service public de l'eau potable en Guadeloupe est plus que jamais préoccupante et elle ne nous fait pas honneur. Il est inacceptable que, en 2021, dans l'un des territoires de la République, nos concitoyens aient des difficultés d'accès à l'eau potable, à cause notamment d'un réseau en mauvais état et d'une gestion désastreuse.

Il est inadmissible qu'un tel degré d'imprévision soit encore possible pour un besoin essentiel. Certes, l'État a pu apporter quelques premières réponses, dans l'urgence. En 2014, le préfet a coordonné l'élaboration d'un plan de sécurisation de l'alimentation en eau potable, lequel fut complété en 2016

Ainsi, le diagnostic auquel il faut répondre n'est que trop simple : la gestion de l'eau potable en Guadeloupe souffre actuellement d'être plurielle et disparate. Au début des années 2010, pas moins de treize entités assuraient l'exercice des compétences « eau potable » et « assainissement Cet éparpillement est la source de désaccords entre les acteurs du service public. En résultent des dysfonctionnements pour les usagers. Il est donc proposé d'instituer un syndicat mixte ouvert, qui regroupera les cinq communautés d'agglomération de Guadeloupe continentale, chacune membre aux côtés du département et de la région. Il s'agit Il s'agit d'une nécessité, même si ce choix nourrit un regret : il implique de contourner le principe de libre administration des collectivités territoriales, en passant par la loi. Toutefois, certains ajustements apportés au texte, notamment par notre rapporteure, devraient permettre d'assouplir le dispositif, afin que celui-ci se rapproche davantage du droit commun des syndicats de gestion de l'eau. Au regard de ces éléments, le syndicat devrait permettre une unification et une mutualisation du service public de l'eau potable. Ainsi, l'on pourra espérer une meilleure gestion, appelée à connaître d'autres améliorations dans les années à venir. le texte que nous examinons crée une commission consultative auprès du syndicat mixte, qui sera chargée de l'organisation des procédures de transparence et d'association des usagers aux mesures prises par le service public de l'eau en Guadeloupe. Nous comptons évidemment sur tous les acteurs de ce dispositif, afin de garantir une gouvernance efficace du syndicat mixte ouvert. Si l'on s'appuie sur les analyses de certains rapports d'expertise, il faudra atteindre progressivement trois objectifs d'abord, être capable, en période normale, d'alimenter en permanence l'ensemble des usagers ; ensuite, être en mesure d'assurer la distribution normale des usagers dans un contexte d'indisponibilité temporaire de la ressource ; enfin, être à même d'assurer l'alimentation en eau face à un aléa exceptionnel.

président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « c'est simple, soit l'eau n'arrive jamais dans nos robinets, soit elle arrive, mais n'est pas potable Ces mots du président du comité de défense des usagers de l'eau en Guadeloupe résument la situation dramatique qui se déroule dans ce territoire. Dans notre République, pour certains l'eau est un « accident

Des rejets toxiques polluent l'eau et menacent la santé des habitants. Rappelons que 90 % des Guadeloupéens ont été empoisonnés par le chlordécone et que la plainte pour mise en danger de la vie d'autrui est menacée de prescription, alors que la toxicité de ce produit est connue depuis les années 1960.

l'accès à cette ressource est reconnu dans notre code de l'environnement et par l'ONU comme un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie.

impose une nouvelle gouvernance face aux échecs des négociations entre élus locaux. Le législateur viendrait créer un syndicat en rendant l'adhésion des collectivités obligatoire. Nous partageons l'ambition de remettre sur pied un service public en faillite et reconnaissons les améliorations apportées pour renforcer le rôle des associations d'usagers. Mais nous regrettons le choix d'imposer cette organisation, qui plus est en passant par la loi. Le consensus local des collectivités et une concertation citoyenne sont essentiels au bon fonctionnement et à la transparence de la structure. Cette intrusion dans l'exercice des compétences peut être vue comme un ultimatum par les Guadeloupéens. nous défendons une conception volontariste des transferts de compétences, conformément à la libre administration des collectivités. Nous craignons surtout que ce cadre législatif ne soit qu'une coquille vide, qu'il ne réponde ni aux défaillances du système de distribution de l'eau ni aux questions soulevées par la création d'un nouveau syndicat. coopération intercommunale, les EPCI, n'est pas réglé, puisque le syndicat se voit transférer la seule dette bancaire : qu'en est-il des dettes fournisseurs ? la remise en état des réseaux de distribution est évalué à près de 1 milliard d'euros. Puisqu'il s'est résigné à s'introduire dans la gestion locale, le Gouvernement aurait pu apporter un soutien financier pour réaliser ces investissements. Le présent texte pose un cadre institutionnel sans apporter de garanties.

le groupe Union Centriste, qui bénéficie de l'expertise de collègues de La Réunion, de Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, connaît bien ce sujet, mais il avait moins eu l'occasion de se poser la question de la situation guadeloupéenne en matière d'eau et d'assainissement. C'est dire si les éléments dont j'ai pris connaissance ont suscité mon étonnement

du rapport de l'Observatoire de l'eau pour 2020. J'avoue avoir découvert avec stupéfaction, dans ce document, que l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, dont la moyenne nationale est 96 sur 120, n'atteint en Guadeloupe que 31 sur 120,

se retrouvent à vivre un quotidien pénible, rythmé par les coupures et les « tours d'eau ». Il est grand temps de garantir à tous un accès continu à l'eau potable

mais aurait opportunément permis d'augmenter les financements de la réhabilitation des réseaux d'eau, pour lesquels chaque euro est crucial. Aussi est-il regrettable que, à l'époque, le Gouvernement, représenté par Mme Girardin,

Ainsi, le 4 mars dernier, les collectivités locales de la Guadeloupe- le conseil départemental, le conseil régional et des EPCI -ont adopté les statuts d'un syndicat mixte ouvert. L'initiative parlementaire est un droit, et la loi est souveraine. Pourtant une question fondamentale, de principes, se pose : la loi doit-elle contraindre les libertés locales ou les protéger ? Nous sommes dans une démocratie ! De plus,

une réponse ambitieuse à la situation de l'eau en Guadeloupe, mais il ne propose pas de régler tous les problèmes. Il fait, en effet, l'impasse sur d'autres points

Ajoutez à cela la réalité financière des collectivités locales de la Guadeloupe, qui nous commande d'appeler, avec lucidité, à un accompagnement massif de l'État. Sans cette aide, comment garantir la viabilité financière de ce projet, sans que les usagers paient au prix fort les investissements à faire sur les réseaux ? Oui, l'État doit prendre ses responsabilités. Comme l'a proposé à maintes reprises notre collègue Victorin Lurel, le Gouvernement devrait accepter de créer des mécanismes exceptionnels de financement des collectivités locales. Plusieurs options sont possibles, passant par le biais du plan de relance, par la création de structures de défaisance, ou, mieux encore, par une garantie d'État, sur trente ans, d'au moins 500 millions d'euros de prêts aux collectivités locales, avec un différé d'amortissement minimal de trois ans. Il s'agit véritablement de reconstruire au plus vite et de manière durable les réseaux d'eau et d'assainissement de la Guadeloupe. Monsieur le ministre, nous sommes toujours dans l'attente d'un engagement tangible de votre part dans cette direction. Les termes et les conditions évoqués dans le contrat de préfiguration que vous avez dicté au président du conseil régional de la Guadeloupe sont sont purement désobligeants envers les élus de la Guadeloupe dans leur ensemble. Nous ne saurions les accepter. La loi doit accompagner et protéger les termes de la discussion locale, non la maîtriser ou la forcer. Nous sommes encore en démocratie Notre volonté est de soutenir les démarches en cours pour assurer au plus tôt l'accès à l'eau potable en Guadeloupe. Je tiens à indiquer que l'État porte une responsabilité

les conditions d'une amélioration durable de la qualité de ces services publics essentiels en Guadeloupe, comme partout ailleurs dans l'Hexagone ou en outre-mer. Or, cela a déjà été souligné par les précédents intervenants, la situation

Celles-ci sont, certes, concentrées dans les régions montagneuses et occidentales de l'île de Basse-Terre, mais cette raison, à elle seule, ne justifie aucunement les difficultés récurrentes du service public de l'eau. la combinaison d'un réseau insuffisamment équipé et entretenu avec l'existence de difficultés de gestion administrative et financière récurrentes a créé une situation inacceptable. Les usagers sont victimes de pénuries ponctuelles, voire de coupures récurrentes, rendues nécessaires pour réguler l'approvisionnement défaillant : les fameux « tours d'eau ». S'y ajoute un prix de l'eau largement supérieur aux moyennes nationales, y compris en comparaison d'autres territoires ultramarins. Cela suscite des impayés, qui fragilisent encore plus la santé financière du système, créant ainsi un cercle vicieux. Cette situation n'a pas seulement pour effet n'a pas seulement pour effet de compliquer la vie quotidienne des Guadeloupéens. Elle crée aussi des perturbations de l'activité économique et constitue une source de risques sanitaires substantiels. Alors que la crise du covid-19 se poursuit et que le CHU de Pointe-à-Pitre se remet encore des suites d'un grave incendie, il est donc important de s'atteler dès que possible à réduire les facteurs de risques dans ce domaine. Il ne revient pas au législateur de débattre des infrastructures à installer ou à rénover dans telle ou telle partie de l'archipel guadeloupéen. Cependant, avant de songer à la réfection de canalisations et à l'installation de pompes, le premier pas pour résoudre le problème semble surtout de rénover le cadre institutionnel. Les tentatives locales pour trouver une solution pérenne n'ont

public local de pilotage du service public de l'eau. Compte tenu de la situation locale que je viens de vous décrire, le présent texte me paraît donc opportun. Le syndicat mixte qu'il crée permettra d'assurer une gouvernance unifiée de l'eau dans la quasi-intégralité du territoire guadeloupéen et sera accompagné d'une commission de surveillance. La commission des lois, sur l'initiative de son rapporteur, notre collègue Françoise Dumont,

à opérer des ajustements au dispositif voté par l'Assemblée nationale. Ces derniers sont destinés à renforcer l'efficacité de la nouvelle structure, par exemple sur la répartition des contributions financières, ou en ce qui concerne la possible future inclusion de l'île de Marie-Galante dans le syndicat.

monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 1 crée une structure unique, un syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement, le 1 septembre prochain. Il s'agit, vous le savez, d'un projet évoqué dès le début de l'année 2015 par le groupe de travail dirigé, à l'époque, par le sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Cette initiative n'a pas prospéré, mais elle a, depuis lors, fait l'objet de nombreux échanges et, surtout, d'un accord de principe entre les élus locaux et les parlementaires guadeloupéens. Les modalités de cette unification n'ont jamais fait consensus, ce qui a privé jusqu'à présent la Guadeloupe d'une nouvelle gouvernance des services publics d'eau et d'assainissement. J'aimerais, par ailleurs, rappeler une évidence cet article n'entrave en rien le principe de la libre administration des collectivités. Il concrétise, au contraire, une initiative commune, qui ne peut rester bloquée indéfiniment. C'est pourquoi il me semble important de préciser que les statuts de ce syndicat seront arrêtés par le préfet après avis des organes délibérants du syndicat mixte ouvert, le SMO, à savoir les cinq communautés d'agglomération de Guadeloupe continentale, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera de Levant, Nord Basse-Terre et CAP Excellence, le conseil départemental et le conseil régional. Le SMO proprement dit sera placé sous la vigilance d'un conseil syndical que nous avons souhaité le plus équilibré et le plus représentatif possible il garantira un meilleur accès à l'eau et à la continuité des services publics d'eau potable et d'assainissement ; il engagera les investissements nécessaires et préservera la ressource ; il assurera, enfin, la gestion de service d'information, de recueil et de traitement des demandes des usagers pour tenter de restaurer une confiance aujourd'hui perdue. Bien sûr, cet article 1 n'entend pas, à lui seul, résoudre l'ensemble des problèmes d'eau et d'assainissement en Guadeloupe, les causes et les facteurs sont trop nombreux, mais nous nous accordons tous sur un fait : il faut un début. Cette structure unique est une première étape, qui nous permettra de reconstruire des services publics à la hauteur des attentes des Guadeloupéens.

Le ministre a bien voulu envoyer un courrier qu'il a présenté comme une feuille de route imposée aux élus, en particulier au président de région, indiquant que son texte n'était « qu'une préfiguration ».

et, singulièrement, depuis 2015. En cela, j'avoue que je comprends l'initiative, même si je désapprouve sa méthode. C'est un peu « en même temps », disons-le, mais je comprends qu'il faille avancer.

à nous abstenir. Je dirai tout à l'heure un petit mot en faveur de la commission des lois, qui a fait un excellent travail de rédaction et de légistique.

d'eau et d'assainissement. Au regard de la gravité de la situation, il me semble relever de la responsabilité du législateur d'agir en procédant à cette unification. Au demeurant, le présent amendement tend à prévoir des modalités particulièrement

Cette proposition, au même titre que l'adhésion facultative au syndicat, ne ferait que prolonger le que la présente proposition de loi entend précisément dépasser. L'entité que nous proposons de créer se doit, en effet, d'être durable et de ne pas dépendre de jeux politiques.

Je ne comprends pas que l'on veuille, si j'ose dire, porter atteinte à la liberté d'un parlementaire de dire ce

sociale de l'eau pour les usagers les plus modestes. Je partage pleinement l'intention des auteurs de cet amendement, le prix de l'eau étant un problème particulièrement aigu en Guadeloupe. J'ai d'ailleurs développé ce point dans mon rapport. Au regard de la situation, l'étude de faisabilité d'une tarification sociale de l'eau semble donc une mesure de bon sens. Je rappelle que l'article 15 de la loi relative à l'engagement dans la vie a pérennisé la possibilité d'une tarification sociale de l'eau. Celle-ci est par ailleurs pleinement applicable au syndicat mixte créé par la présente proposition de loi. Il reviendra donc aux membres du syndicat mixte de s'approprier, une fois sa faisabilité étudiée, cette possibilité.

est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à prévoir en effet que deux représentants d'usagers et deux personnalités qualifiées siègent au sein du comité syndical. Or un tel ajout pose trois difficultés. d'abord, il nuit à la lisibilité et à la cohérence de la gouvernance du syndicat mixte. Les usagers et personnalités qualifiées qui sont représentés au sein de la commission de surveillance pourraient voir leur rôle de contrôle au sein de cette commission brouillé par une telle disposition. Ensuite, il pose une difficulté juridique, en ce qu'il associerait à la direction d'un syndicat mixte des personnalités qui n'en sont pas membres. Or un syndicat mixte a vocation à agir en fonction des choix de ses membres. Enfin, sur le plan technique, le présent amendement ne vise à prévoir aucune procédure de nomination de ces personnalités qualifiées

supprimer la présence des personnalités qualifiées et des représentants d'usagers dans le comité de surveillance.

a été rejeté en commission. La modification proposée me semble au surplus excessive et problématique sur le plan juridique. Par définition, le comité syndical, qui a la charge de l'administration du syndicat mixte unique, doit être composé de délégués des membres. l'avis du Gouvernement ?

est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à octroyer quatre sièges à la commission de surveillance au sein du comité syndical. J'en comprends certes l'intention, mais il me semble inopportun. La gouvernance du syndicat, telle qu'elle résulte de la rédaction actuelle de la proposition de loi, est claire : le comité syndical administre la commission de surveillance et la commission de surveillance contrôle ses actes. Placer des représentants auprès du comité syndical brouillerait cette gouvernance en la mettant en situation d'être à la fois juge et partie. Comment contrôler efficacement un organe que l'on contribue à diriger ? Il semble préférable de conserver une répartition des tâches bien établie. Je rappelle, au surplus, que la commission des lois a renforcé le rôle de la commission de surveillance en prévoyant une procédure d'audition réciproque par le comité syndical et la commission de surveillance. Par ailleurs, un tel ajout au comité syndical serait déséquilibré sur le plan juridique. Un syndicat mixte ne doit être administré au sein du comité syndical que par ses membres. Ouvrir davantage cet organe de direction semble donc particulièrement problématique

proportionnellement à leur population. Le texte, tel qu'il est rédigé, prévoit déjà qu'une telle répartition s'effectue proportionnellement au nombre d'usagers situés sur le territoire de chaque EPCI.

sur la soutenabilité financière et économique de la structure unique et son impact sur le coût de l'eau en Guadeloupe. Je comprends, naturellement, l'importance des sujets financiers pour la pérennité de la structure nouvellement créée. Néanmoins, conformément à une position constante de la commission des lois et du Sénat, les demandes de rapport sont systématiquement rejetées. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j'émettrais un avis défavorable.

est à M. Dominique Théophile, sur l'article. La défaillance des services publics d'eau et d'assainissement et l'institutionnalisation de ce que l'on appelle les « tours d'eau » sont à l'origine de la défiance des Guadeloupéens. C'est ce qu'a pu constater Mme la rapporteure lorsqu'elle a auditionné pas moins de dix associations et collectifs d'usagers. Face à ce climat de défiance, l'article 2 tend à créer une commission de surveillance placée auprès du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. Celle-ci sera composée des usagers du service public, des représentants des membres du SMO, des représentants de la de la chambre d'agriculture, de la chambre de métiers et de l'artisanat, du président de l'association des maires de Guadeloupe et des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences. Elle sera présidée par un président des associations d'usagers, sera chargée de veiller à la transparence des services publics d'eau et d'assainissement et associera les usagers aux mesures qui seront prises. Le contrôle de la commission de surveillance par les représentants des associations d'usagers est donc doublement garanti. Tout d'abord, parce que la moitié des sièges leur sera réservée. Ensuite, parce que la présidence de la commission leur reviendra, auront ainsi une voix prépondérante en cas d'égalité de vote. Cette proposition suit ainsi les préconisations des rapports et des audits menés sur ce sujet et pose les bases d'une nouvelle gouvernance plus transparente et responsable devant les usagers.

Cet amendement vise à clarifier la procédure de nomination à la commission de surveillance sur proposition du représentant de l'État en Guadeloupe, après avis, en fonction des membres, soit du président du syndicat mixte, soit des chambres consulaires de Guadeloupe, soit de l'association des maires de Guadeloupe. Pour ce faire, il tend à prévoir les modalités de transmission de l'avis au préfet par les personnes consultées sur la proposition de nomination. Ces dernières disposeront d'un délai d'un mois afin de rendre par écrit leur avis au préfet. À défaut, celui-ci sera réputé favorable, afin de ne pas paralyser les procédures de nomination à la commission de surveillance.

de la commission de surveillance. La commission des lois a précisé la procédure d'inscription à l'ordre du jour du comité syndical d'une question de la commission de surveillance en trouvant ainsi un nouvel équilibre. Si cette question doit avoir un lien avec l'ordre du jour, elle peut désormais être inscrite à la demande de la majorité des membres ou sur proposition du seul président de la commission. M. Benarroche souhaite aller plus loin et imposer l'inscription d'une question dès la deuxième demande par la commission de surveillance. Il me semble difficile d'adopter un tel amendement, dès lors que celui-ci tend à figer la procédure de sollicitation engorger l'ordre du jour du comité syndical. Je propose de nous en tenir à la voie médiane trouvée par la commission, c'est-à-dire à une possibilité d'inscription à l'ordre du jour, en parallèle d'une possibilité d'émettre des avis et propositions sur tout sujet relevant de la compétence du syndicat mixte. La commission émet donc un avis défavorable

du syndicat mixte. Cela permettra, me semble-t-il, de renforcer l'information des associations d'usagers sur les finances de ce syndicat et de parfaire leur contrôle. La commission émet

ayant commis des manquements reversent les rémunérations indûment perçues. Cet amendement me semble néanmoins inopportun. Premièrement, son objet semble relever davantage de la compétence du juge que de celle du législateur. Il ne revient ainsi pas à ce dernier de se prononcer sur la nature des manquements avérés mentionnés, pas plus que sur l'étendue des rémunérations indûment perçues. Si les personnes publiques attributaires de la compétence et délégantes se considéraient lésées dans les modalités d'exécution des contrats passés avec les entreprises délégataires, il leur reviendrait de saisir le juge administratif. Deuxièmement, l'amendement semble juridiquement problématique et dépourvu d'effets concrets, faute de prévoir une procédure précise de recouvrement des sommes concernées. Par ailleurs, une telle disposition placerait le syndicat mixte unique nouvellement créé dans la position de réclamer des sommes à des délégataires avec lesquels il n'a jamais contracté, les cocontractants étant les EPCI exerçant aujourd'hui la compétence. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable Monsieur le ministre, tel était le cas, il faudrait contrôler l'action du Gouvernement pour que les instructions soient données dans le bon sens. Vous dites qu'il y a eu des carences de l'État au niveau du contrôle de légalité. Ce n'est pas exact. Certes, il y a eu des carences de l'État

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur l'article 36 de notre règlement. Le Gouvernement a demandé, hier, que la suite de l'examen de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école soit inscrite à l'ordre du jour de ce mercredi 10 mars, à l'issue de l'espace réservé au groupe RDPI, et éventuellement le soir, en vertu de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution. Cette initiative inédite, me semble-t-il, pose question. Nous demandons que l'article 48 de la Constitution soit examiné avec la plus grande précision. Son alinéa 3 donne un grand pouvoir au Gouvernement pour enclencher l'ordre du jour prioritaire, mais son alinéa 4 accorde une compétence exclusive à l'assemblée concernée pour organiser l'ordre du jour des séances consacrées à l'initiative parlementaire, dit « ordre du jour réservé ». Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée, à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée, ainsi qu'à celle des groupes minoritaires. La conférence des présidents a fait le choix de ne pas recourir à la soirée de ce jour de séance réservée à l'initiative parlementaire. Ce n'est pas pour autant que le Gouvernement peut l'utiliser à sa guise. L'alinéa 4 l'interdit même expressément. Par ailleurs, nous estimons que cette intervention du Gouvernement rompt l'égalité de traitement entre les groupes. En effet, ceux qui ne soutiennent pas le Gouvernement ont un espace limité à quatre

a déjà trop souvent pris l'habitude d'utiliser les propositions de loi, non soumises à l'avis du Conseil d'État et dépourvues d'étude d'impact, comme véhicules législatifs. Aujourd'hui, il en vient à utiliser les espaces réservés aux groupes

! Nous demandons également l'application stricte de l'article 48, alinéa 4 de la Constitution. Acte vous est

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux que soit présentée aujourd'hui au Sénat la proposition de loi de Mme la députée Cécile Rilhac. Cette proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école est l'occasion pour moi de rappeler une nouvelle fois, devant la représentation nationale, l'engagement remarquable de ces directeurs depuis le début de la crise sanitaire. Si nous pouvons afficher aujourd'hui une maîtrise des chaînes de contamination dans les écoles, et ce depuis plusieurs mois, avec un nombre de cas de contamination stable et un nombre très bas de fermetures de classes et d'écoles, ciblées par territoire,

Ce sont eux aussi qui, depuis septembre, veillent à l'application de l'ensemble des mesures sanitaires et mettent en oeuvre les mesures d'accompagnement personnalisé qui s'imposent pour beaucoup d'élèves. Il y aurait mille et un exemples à donner de l'ampleur de leur travail et de leur engagement de chaque jour. Les parents d'élèves le savent, qui les voient agir au quotidien. D'année en année, les missions et les responsabilités des directrices et directeurs d'école se sont considérablement accrues. Aujourd'hui plus qu'hier, ils doivent dialoguer avec les parents d'élèves, les collectivités, porter le cadre de l'institution et le garantir, accompagner les évaluations nationales et les évolutions pédagogiques. les évolutions pédagogiques. Ces évolutions exigent des compétences plus importantes au quotidien, un positionnement plus fort dans notre institution, des responsabilités plus grandes et mieux reconnues. Ces évolutions sont nécessaires. Et cette conviction, mesdames, messieurs les sénateurs, a toujours été la mienne. Depuis mon arrivée au Gouvernement, vous le savez, j'ai fait de l'école primaire la priorité de mon ministère.

Dès l'été 2019, j'ai souhaité que le chantier de l'amélioration de la situation des directrices et des directeurs d'école fasse partie de l'agenda social du ministère. Comme vous le savez, nous avons ainsi conduit une phase de diagnostic qui a reposé, pour partie, sur une consultation en ligne à laquelle les deux tiers des directeurs ont répondu. Nous avons rendu publics les résultats de cette consultation, qui nous a permis de mesurer l'ampleur de l'attente de nos directrices et directeurs d'école. Les travaux ont été engagés, et les premières réponses ont été apportées. Depuis septembre dernier, en effet, plusieurs évolutions permettent d'améliorer l'exercice de leurs missions. J'en évoquerai les principales. En premier lieu, afin de leur donner plus d'autonomie dans l'exercice de leur métier et d'alléger leurs tâches administratives, j'ai souhaité qu'ils aient la pleine responsabilité de la programmation et de la mise en oeuvre des 108 heures annuelles de service dans le cadre réglementaire existant. Cette mesure s'est accompagnée d'une rationalisation du nombre et du calendrier des enquêtes, ainsi que d'une recherche d'amélioration de leurs outils numériques de gestion. Tout cela contribue à alléger le carcan administratif et à redonner aux directeurs d'école les marges de manoeuvre nécessaires, pour leur permettre de se recentrer sur l'essentiel, à savoir le pilotage de leur école.

S'y ajoutent 900 nouveaux contrats de préprofessionnalisation signés ou en cours de signature. Ces contrats permettent à des jeunes qui se destinent au métier de professeur de s'y préparer, tout en renforçant les capacités d'encadrement de l'école. En complément de ces appuis précieux, sinon indispensables, et dans l'attente du vote de la proposition de loi, nous expérimentons depuis la dernière rentrée une fonction de référent pour les directrices et directeurs d'école. Placés auprès des directions des services départementaux de l'éducation nationale, ces référents leur apportent écoute et conseils dans l'exercice de leurs missions. Cet accompagnement vient compléter les deux journées de formation minimum désormais accordées aux directrices et directeurs.

À la rentrée de 2021, comme je m'y étais engagé, un nouveau régime des décharges sera installé. J'ai d'ores et déjà annoncé que 600 emplois supplémentaires seraient consacrés au renforcement des décharges des directrices et directeurs d'école, leur répartition ayant fait l'objet d'une large concertation avec les organisations représentatives. Enfin, en ce moment même, nous travaillons avec les partenaires sociaux sur la possibilité d'une délégation de compétences des inspecteurs de l'éducation nationale. Comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, j'y suis favorable ; nous en reparlerons sans doute. Les directeurs bénéficieraient alors de marges de manoeuvre beaucoup plus grandes, dans une juste adéquation avec leur niveau de responsabilité réel.

Je veux croire que cet exposé vous aura montré combien notre ministère a pris à bras-le-corps cette question, dont les enjeux sont intimement liés à la réussite de nos élèves. L'étape d'aujourd'hui est très importante. La proposition de loi de Mme la députée Cécile Rilhac, que je salue, a pour objet de consacrer, sinon de renforcer, par la loi la plupart des mesures que je viens de vous présenter, qu'il s'agisse de la reconnaissance nécessaire de la fonction de directrice ou directeur d'école, de l'autonomie de ces professionnels, de l'accompagnement matériel et humain auquel ils pourront prétendre et du nouveau régime de décharges dont ils bénéficieront.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,d'un côté, « polyvalence », « responsabilité », « sens du relationnel », « tâches administratives », « disponibilité

Les 45 000 directrices et directeurs d'école de notre pays sont un maillon essentiel du bon fonctionnement des écoles. Ils sont des figures identifiées et connues,

que 94 % des directeurs d'école cumulent charge de classe et direction d'école ; seuls 6 % d'entre eux sont entièrement déchargés. La poursuite de la pandémie, avec l'évolution des protocoles sanitaires, la gestion des suspicions de covid et des cas de covid avérés continuent de souligner l'ampleur de leurs responsabilités. Cette crise met en lumière le changement des missions des directeurs d'école du fait de l'évolution de la société, de la modification des relations entre les parents et l'école, ou encore du développement de l'école inclusive, dont nous nous réjouissons. si les responsabilités ont augmenté, les textes juridiques, eux, n'ont pas évolué. Le juridique, administratif et humain est devenu intenable. La commission de la culture, au travers du rapport très juste de nos collègues Max Brisson et Françoise Laborde, avait identifié les cinq besoins des directeurs d'école

Nous vivons un moment de convergence : un rapport du Sénat dénonçant un intenable ; une proposition de loi de nos collègues députés

Tels sont les objectifs de cette proposition de loi que le Sénat peut adopter aujourd'hui. J'espère que nous aurons un débat riche sur le fond. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi créant la fonction de directrice et directeur d'école a été déposée à l'Assemblée nationale en mai 2020 dans un contexte très particulier. Le 29 septembre 2019, Christine Renon s'est suicidée dans son école de Pantin. Les courriers qu'elle avait adressés à ses collègues, ainsi qu'à l'éducation nationale, ont fait ressortir le malaise grandissant des directrices et directeurs d'école. Le constat est simple. Les directrices et directeurs dénoncent un manque de reconnaissance, une charge de travail trop lourde, avec trop peu de décharges de classe et quasiment aucune aide administrative, ainsi qu'un manque de revalorisation salariale. En 2018, selon le rapport d'information de la commission de la culture du Sénat présenté par Max Brisson et Françoise Laborde, près de 60 % d'entre eux déclaraient être en situation de burn-out. La fonction de directrice et directeur d'école attire de moins en moins les enseignants, car elle relève davantage d'un sacerdoce que d'une promotion valorisante. D'ailleurs, selon les syndicats, près de 4 000 postes de directeur seraient vacants, ce qui représente 9 % des écoles. Face à cette situation, peu de choses ont été faites, monsieur le ministre, à part le dépôt de cette proposition de loi par la députée de votre majorité Cécile Rilhac. Vous avez ensuite lancé, en décembre 2019, une grande consultation des directrices et directeurs d'école, qui ont été très nombreux à répondre. Les résultats sont parlants : quelque 75 % d'entre eux consacrent une grande partie de leur temps aux tâches administratives, et 62 % disent que ces tâches sont les plus pénibles. Vous avez concédé une augmentation de 600 postes destinés aux décharges de direction, ainsi qu'une prime de 450 euros brut par an, dont vous avez annoncé qu'elle serait pérennisée. C'est malheureusement bien loin d'être suffisant ! Et que représentent 600 postes, alors que la France compte plus de 44 000 écoles publiques et qu'une majorité de leurs directeurs disent manquer de temps Le contexte s'est aggravé en 2020 avec la période inédite de la crise sanitaire, qui a placé les équipes enseignantes dans un environnement dégradé. Celles-ci ont été, et sont toujours, particulièrement exposées. Elles font face à l'isolement et à une charge de responsabilité accrue. Je tiens aujourd'hui à les féliciter, à leur rendre hommage et à souligner leur professionnalisme à toute épreuve et leur engagement sans faille. Quelles sont les demandes ? Les directrices et directeurs d'école veulent une aide administrative pérenne, assurée par des permanents et non par des jeunes en service civique, qui changent tous les ans et ont besoin d'être formés à chaque rentrée.

Certes, pour le moment, la création d'un emploi fonctionnel a été retirée du texte à l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose. Mais cette proposition va revenir. Nous tenons à saluer la volonté de reconnaître et d'augmenter les possibilités de décharge, mais il faudrait clarifier Le risque de créer une hiérarchie entre le directeur et les enseignants est toujours présent. Les syndicats et la majorité des enseignants que nous avons interrogés s'accordent pourtant sur ce point : il faut conserver le fonctionnement collégial des écoles. De plus, différentes mesures laissent craindre une augmentation de la charge de travail des directrices et directeurs, notamment la création d'une mission de formation, ce qui va à contresens de leurs demandes. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne votera donc pas cette proposition de loi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « surcharge de travail administratif », « manque de reconnaissance », « solitude » : les directeurs et directrices d'école expriment bien souvent par ces mots les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Dans un rapport d'information de grande qualité, notre collègue Max Brisson et notre chère Françoise Laborde ont présenté de nombreux témoignages illustrant cette réalité, qui n'est pas sans conséquence sur les vocations. Chaque année, ce sont en effet près de 4 000 postes de directeur qui restent vacants. Le rôle de directeur d'école est pourtant essentiel au fonctionnement de l'école au regard des nombreuses missions qu'il occupe. Je ne vais pas les énumérer, car cela a été fait. Je rappellerai seulement que ces missions se sont progressivement renforcées au gré des défis auxquels notre société est confrontée. La pandémie actuelle en fait partie. Plus que jamais, ce grand défi sanitaire a mis en lumière la mobilisation extraordinaire des directions scolaires. En 2020, le Gouvernement a accéléré l'agenda social, avec la nécessité impérieuse de soutenir cette catégorie. Le texte qui nous est proposé va dans ce sens. On y retrouve de nombreuses propositions du rapport du Sénat que j'ai évoqué au début de mon propos. Oui, il est nécessaire de reconnaître, à l'article 2, que le directeur dispose d'un emploi de direction et que doivent être attachées à ce rôle des gratifications à la hauteur de son investissement et de la grande disponibilité qu'impliquent ses missions croissantes. En effet, presque tous les directeurs et directrices dépassent leur temps de travail hebdomadaire. Au-delà de leur statut, les directeurs réclament aussi davantage de moyens humains pour faire fonctionner l'école. La mise en place d'une assistance administrative et matérielle, prévue par l'article 2 , est une bonne chose. Toutefois, il faut faire attention à ne pas trop solliciter les collectivités locales. Ce ne sont pas nos communes et nos départements qui alourdissent les charges incombant aux directeurs. en particulier assumer les nouvelles responsabilités qu'il impose aux directeurs au travers de ses politiques nationales. Je pense aux plans de sécurité renforcés depuis les attentats de 2015, mais aussi au développement de l'école inclusive. Bien entendu, on ne peut que souscrire au développement de ces politiques fondamentales, mais les moyens doivent suivre sur le terrain. L'article 1, qui octroie une délégation de compétences de l'autorité académique aux directeurs, est également une avancée, que mon groupe partage. Le directeur a besoin d'une respiration pour prendre des initiatives sans devoir toujours se justifier. Cependant, j'observe que, à ce niveau du texte, se pose la question de l'autorité fonctionnelle. Au vu des amendements déposés, ce point va faire débat. Est-il utile, comme l'ont fait les députés en première lecture, de préciser que le directeur n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants de son école ? La commission a supprimé cette mention. Il faut en effet trouver un équilibre qui ne remette pas en question la place de chacun dans l'école. L'indépendance des professeurs et leur liberté pédagogique sont consubstantielles à notre système éducatif. le directeur doit avoir les moyens de son rôle, car il s'est progressivement transformé en un véritable chef d'établissement. Mes chers collègues, le groupe du RDSE aborde ce texte avec bienveillance, mais il faudra sans doute faire encore plus, car l'école de Jules Ferry a bien changé. Sur certains territoires, elle est devenue le réceptacle de nombreuses fractures sociales que les directeurs et directrices tentent de colmater avec leur énergie, leur temps et leur humanité. Ceux-ci méritent à ce titre notre admiration et, surtout, tout notre soutien pour leur large contribution au pacte républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mal-être des directeurs et des directrices d'école est connu, tout comme l'est leur surcharge de travail, particulièrement en ces temps d'épidémie.

Vous avez annoncé, monsieur le ministre, quelques avancées bienvenues : je pense aux décharges, par exemple, en regrettant que ces dernières ne concernent qu'une minorité des directeurs et directrices d'école, qui se voient confier en parallèle de nouvelles missions. Les postes qui sont créés pour compenser cette mesure sont très insuffisants, alors que l'on manque déjà tellement de remplaçants. La pérennisation de la prime exceptionnelle de 450 euros est une bonne nouvelle, même si elle est encore loin de permettre de rattraper les écarts de rémunération avec les autres pays de l'OCDE. Depuis des années, les tâches administratives des directeurs et directrices d'école augmentent sans qu'une aide efficace leur soit apportée, et ce n'est évidemment pas les jeunes en service civique qui pourront y répondre. Ce problème se pose avec plus de force encore en ces temps de crise sanitaire, où la mise en oeuvre de protocoles, les injonctions parfois contradictoires et les délais contraints pèsent jusqu'à l'épuisement. Les directeurs et les directrices sont au croisement des exigences des parents, des enseignants, des autorités académiques et parfois des communes ; et le soutien hiérarchique leur manque quelquefois cruellement.

J'en viens à ce qui sera sûrement un point de discussion majeur de la proposition de loi : la place qu'occupent les directeurs et les directrices d'école maternelle et élémentaire dans l'organisation scolaire. Il y a un an, une directrice d'école déclarait à notre commission : « Pour être efficaces, nous avons besoin de continuer à être enseignants. Notre voix sera plus forte si nous vivons les mêmes problèmes que nos collègues. » Il faut entendre cette volonté, tenir compte de la consultation que vous avez lancée, monsieur le ministre, et dont la conclusion est la même. En effet, la crainte est grande d'aller vers des directeurs uniquement gestionnaires, comme le deviennent parfois les principaux de collèges et les proviseurs de lycées,

Cette nouvelle offensive pour modifier le statut des directeurs d'école intervient en même temps que des pressions fortes pour regrouper les écoles de proximité dans de super-établissements. Comment ne pas faire le lien ? Pendant la crise, c'est le collectif qui a permis que les écoles tiennent, m'ont expliqué des directeurs et des directrices d'école. Ni l'autorité hiérarchique ni le concept quelque peu « fumeux »- vous m'excuserez, mes chers collègues, de ce qualificatif -d'« autorité fonctionnelle fonctionnelle » ne permettront d'améliorer la situation de ces fonctionnaires, actuellement débordés, qui demandent du soutien, de l'assistance administrative, de la reconnaissance à tous points de vue, des outils modernes et efficaces, et non pas d'être soumis à davantage de responsabilités dans un contexte déjà difficile, ce qui risquerait au contraire d'accroître la crise de recrutement. Dernier point, plusieurs aspects de ce texte sont inquiétants pour les communes. Celles-ci risquent d'être sollicitées plus encore pour assurer le fonctionnement et la mise à disposition de personnels et de moyens pour les écoles. Ce n'est pas juste sur le fond et, là encore, ce n'est vraiment pas le moment, alors qu'elles ont toutes dû déployer bien des moyens pour faire face à la crise sanitaire et assurer la mise en oeuvre des protocoles. Notre groupe ne soutiendra pas ce texte.

la crise sanitaire a renforcé de manière indéniable le rôle primordial des directeurs d'école. Ceux-ci ont en effet été les piliers, avec les enseignants, de la continuité pédagogique, mettant en place en urgence des outils numériques, organisant l'accueil des enfants du personnel soignant et maintenant le lien entre les enseignants, les parents, les élèves et les mairies.

Au-delà de cette crise, les directrices et directeurs sont bien un maillon essentiel du bon fonctionnement des écoles, dans leur dimension sociale et sociétale : ils sont les interlocuteurs de la hiérarchie académique, des élus locaux et des services municipaux, et des familles. Ils sont aussi membres à part entière de l'équipe éducative, quand ils enseignent encore. Ces constats sont un hommage qui est rendu à ces directrices et directeurs ; mais, en creux, ils mettent aussi en lumière toutes les missions qui leur incombent : ils sont, pour utiliser une expression certes prosaïque, de véritables « couteaux suisses » de l'école de la République sur le terrain. En effet, l'évolution de la société et de l'école a conduit à un renforcement de leurs responsabilités, à une complexification de leurs tâches et à une augmentation du temps qu'ils doivent consacrer à celles-ci. Or, le cadre législatif de leur action n'a pas connu de modifications majeures depuis 2005. Dans leur rapport remis en juin dernier, nos collègues Max Brisson et Françoise Laborde avaient fait plusieurs constats. Tout d'abord, ils avaient rappelé que la fonction de directeur attire moins. Entre 4 000 et 5 000 postes de directeurs seraient vacants chaque année, soit 9 % des écoles, et 13 % des directeurs d'école indiquaient ne pas avoir demandé à exercer cette fonction, ce phénomène touchant les écoles rurales comme les plus grosses structures urbaines. Ensuite, ils avaient relevé que la profession était marquée par un profond malaise. En 2018, plus de la moitié des directeurs d'école considérait que leurs conditions de travail s'étaient dégradées ces dernières années. Ces dégradations mènent parfois à des drames humains, que l'on a tous tristement en mémoire. Le étant devenu intenable, il était vital que l'emploi de directrice ou de directeur soit traité de manière autonome. Le texte qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une volonté commune du législateur et de l'exécutif celle d'améliorer la situation et la reconnaissance des directeurs d'école. Le travail effectué par le rapporteur, Julien Bargeton, a vraiment permis d'aller en ce sens. Le premier point du texte que je souhaite aborder est celui de l'autorité du directeur sur les enseignants. pair parmi ses pairs », comme le veut la formule consacrée. La question de l'autorité hiérarchique doit être évacuée : nombreux sont ceux qui préfèrent une autorité fonctionnelle, car elle évite, entre autres, l'écueil des évaluations des collègues. Nous avons donc souhaité déposer un amendement en ce sens. L'autorité fonctionnelle pour les directeurs favorise le bon fonctionnement de l'école et permet la réalisation des missions qui leur sont confiées c'est une délégation de compétence de l'autorité administrative. En dehors de ce rôle, il n'y a pas d'autorité hiérarchique nécessaire : l'autorité est donc confiée dans les limites du cadre de leur mission. C'est la reconnaissance aussi que l'emploi de directeur d'école est un sujet à part entière

En effet, le texte de l'Assemblée nationale ne prévoit que des raisons structurelles pour déterminer la décharge, à savoir le nombre de classes et les spécificités de l'école. Ces motifs sont trop théoriques et trop rigides. Il existe en pratique des situations imprévisibles, conjoncturelles, qui échappent à l'arithmétique pure et nécessitent l'utilisation d'heures de décharge : prises en charge de handicaps complexes, conflits internes par exemple. Le temps qui leur est consacré peut déborder largement le cadre de la décharge initialement prévue. Un autre point important est celui de la formation. L'article 2 de la proposition de loi pourra être complété lors de notre débat par l'inscription de la nécessité d'une formation initiale sur le rôle, les responsabilités et les missions du directeur d'école, ainsi que par une formation continue adaptée une fois en fonction. En effet, les auditions ont montré que le besoin est réel, notamment en matière de gestion de crise, d'animation et de pilotage. Enfin, le financement de l'accompagnement administratif et matériel à l'exercice de direction pose question. L'État ne doit pas laisser la charge financière peser uniquement sur les communes et leurs groupements. Nous avons donc souhaité déposer un amendement visant à ce que l'État prenne à sa charge ce financement. Toutes les communes n'ont pas les moyens d'assurer aux directeurs d'école un appui technique et humain en matière administrative.

que nous ayons ainsi l'occasion d'évoquer la situation de ces femmes et de ces hommes qui sont des rouages indispensables de nos écoles du premier degré, encore mis à l'épreuve par la gestion récente de la crise sanitaire. La disparition tragique en 2019 de Christine Renon, directrice d'école à Pantin, avait jeté une lumière crue sur une réalité trop longtemps ignorée : accumulation des tâches administratives jusqu'à l'épuisement, carences matérielles, turnover incessant des remplaçants, accompagnement insuffisant de l'académie. Autant de points sur lesquels l'éducation nationale peut et doit s'améliorer, particulièrement dans ses pratiques quotidiennes. Alors que nous étions mobilisés lundi autour de la journée du 8 mars, je souhaite rappeler que 71 % des postes de direction d'école sont occupés par des femmes, majoritaires comme dans bien d'autres champs de l'éducation nationale. Il est plus que temps de reconnaître à leur juste valeur leur travail et leur engagement. Si nous nous rejoignons toutes et tous sur la nécessité de mieux reconnaître et valoriser les directeurs et directrices d'école dans l'exercice de leurs missions, nous différons en revanche sur la meilleure façon d'y parvenir. Les directeurs et directrices d'école n'ont de cesse de dire qu'ils manquent avant tout de temps de décharge, d'aide administrative et de formation. Nous estimons, au sein du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, que c'est par de tels leviers que nous pourrons répondre à leurs attentes, et non par l'affirmation d'une position d'autorité, dont ils ne sont pas demandeurs, L'école du premier degré s'inscrit en effet dans une vision collective incarnée par le conseil des maîtres, dont fait partie le directeur ou la directrice d'école. Son appartenance au corps enseignant est un atout, car elle constitue un gage de sa bonne compréhension des ressorts du métier. Les amendements que nous avons déposés sur l'article 1 de cette proposition de loi qui vise à délimiter le rôle du directeur d'école tendent à réaffirmer cette vision, en énonçant explicitement que le directeur d'école n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants de son école et en délimitant la portée de la délégation de compétences par l'inspecteur d'académie. Les directeurs ne souhaitent pas non plus que leur soient dévolues de nouvelles missions ne relevant pas du cadre actuel de leur fonction. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement de retrait de la mention des « missions de formation » évoquées à l'article 2. Nous avons souhaité préciser dans ce même article 2, qui traite de la fonction des directeurs d'école, le rôle du directeur en matière de projet pédagogique. Nous aurions aimé profiter de l'examen de cette proposition de loi pour faire avancer concrètement les conditions matérielles d'exercice de la fonction de directeur, notamment sur la question des décharges. Nous sommes malheureusement freinés dans cette ambition par l'article 40 Il est cependant essentiel d'affirmer l'importance de ces temps de décharge et la nécessité de garantir qu'ils sont bien ouverts et effectifs pour l'ensemble des directeurs. L'aide administrative est une autre question charnière pour les directeurs d'école. Nous regrettons, à ce titre, la formulation ambiguë de l'article 2 , qui comporte le risque d'entraîner un désengagement de l'État en la matière. Nous saluons en revanche la création d'un « référent direction d'école » dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale introduite par l'article 3. espérons que ce nouvel interlocuteur sera en mesure de jouer un rôle d'appui auprès des directeurs qui font état d'une certaine solitude dans l'exercice de leurs missions. Nous ne saurions trop insister sur la nécessité de circonscrire le cadre de ces missions et de ne pas alourdir la charge de travail des directeurs par de nouvelles prérogatives. À cet égard, la possibilité, prévue à l'article 4, pour les directeurs et directrices d'être chargés de l'organisation du temps périscolaire nous paraît nous paraît ouvrir une brèche dangereuse, alors que cette organisation revient aujourd'hui aux collectivités qui les financent. Le texte suspend certes cette possibilité au consentement du directeur, mais il est facile d'imaginer un scénario où il se retrouverait contraint d'endosser cette responsabilité, sans même évoquer les difficultés matérielles et juridiques soulevées par une telle évolution. Les collectivités, qui financent ce temps périscolaire, sont aguerries à cette organisation qui relève d'abord d'une question de gestion de personnels. C'est la raison pour laquelle nous défendrons la suppression de cet article. Nous ferons par ailleurs preuve de prudence quant à la possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, pour le directeur d'école de recourir à un scrutin par voie électronique lors des élections des représentants des parents d'élèves. Si cette modalité d'organisation apparaît souhaitable, nous devons en effet nous poser la question de l'accès de l'ensemble des parents à un tel scrutin, d'autant que la crise sanitaire nous a démontré à quel point la fracture numérique demeure vivace.

Vous l'aurez compris, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain salue quelques petites avancées introduites par ce texte ; en revanche, il reste très dubitatif sur sa capacité à répondre dans son ensemble aux nombreuses attentes.

L'école est un creuset républicain, un vecteur d'émancipation pour l'ensemble de notre société. Soutenons les directeurs et directrices, qui en sont le coeur battant, et offrons-leur des moyens à la hauteur de cette ambition

pour « mettre fin à un intenable, celui de directeur d'école ». Ces propositions étaient adoptées par notre commission en juin 2020, au moment même où la proposition de loi qui nous rassemble ce jour était déposée à l'Assemblée nationale par notre collègue Cécile Rilhac, que je salue en tribune. Hasard du calendrier, nos travaux se sont croisés, et loin d'en prendre ombrage, je crois que cette volonté commune d'améliorer la situation des directeurs d'école crée des conditions favorables pour répondre à leurs nombreuses attentes. attentes. Dans ce contexte, je veux saluer également les travaux de notre rapporteur, Julien Bargeton, qui nous ont permis de mieux cerner encore les points de convergence qui émergent, ainsi que les éléments dont nous avons encore à débattre. encore à débattre. Tout le monde est d'accord pour dire que sur les directeurs d'école reposent des charges croissantes, de plus en plus complexes. Ces charges proviennent d'une administration toujours plus demanderesse de rapports, de statistiques et d'évaluations. Elles proviennent également de parents de plus en plus exigeants, qui attendent toujours davantage d'une institution dont le directeur est, comme le maire, « à portée d'engueulade », pour reprendre l'expression du président Larcher. Enfin, ces charges croissantes sont amplifiées par les règles et protocoles, toujours plus nombreux à mettre en oeuvre, dans un contexte sécuritaire et sanitaire de plus en plus anxiogène. Face à ces charges croissantes, les directeurs réclament, depuis bien longtemps, plus de temps pour exercer leurs missions. Ils demandent aussi plus d'aide administrative, alors que les contrats aidés ont disparu et que le numérique, loin d'avoir réduit la soif des remontées en tout genre, l'a au contraire amplifiée.

Si personne ne demande un statut et encore moins la création d'un corps, beaucoup souhaitent que l'emploi de directeur soit reconnu comme un emploi fonctionnel, nécessitant davantage de temps et de moyens. Mes chers collègues, voilà ce qui fait consensus ; il est grand temps d'y donner corps. si le suicide de Christine Renon a permis l'émergence d'une prise de conscience et si les données chiffrées portant sur le moral des directeurs d'école nous renseignent sur l'ampleur du malaise-

qui établit enfin, dans le code de l'éducation, que le directeur d'école occupe un emploi de direction, doté d'une délégation de compétences de l'autorité académique. En un mot, mes chers collègues,

Certes, donner une autorité hiérarchique à un jeune directeur d'une école de deux ou trois classes n'a pas grand sens, j'en conviens. Mais en va-t-il de même lorsque l'école compte vingt classes ou plus et près de 450 élèves et que son directeur est déchargé de tout enseignement ? Tout le monde s'accorde à le dire, dans cette situation, celui qui exerce cette responsabilité doit pouvoir disposer des moyens et de la formation nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Tel est le sens des amendements que le groupe Les Républicains a déposés.

Mes chers collègues, je mesure combien nous touchons à un sujet sensible. Je mesure également à quel point les attentes des directeurs d'école sont vives et combien nous devons trouver le point d'équilibre. Nous y réussirons en refusant toute position dogmatique, coupée du fonctionnement quotidien réel de nos écoles, dont nous avons déjà eu quelques belles illustrations précédemment. C'est de cette manière que le groupe Les Républicains appréhende l'examen de cette proposition de loi, qui est

cette proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école était très attendue. À la fois responsables du pilotage pédagogique et du fonctionnement de l'école, tout en jouant un rôle de facilitateurs entre les différents acteurs, les directeurs d'école connaissent une forte augmentation de leurs responsabilités et de leur charge de travail. Pourtant, leur mission reste peu valorisée et, par voie de conséquence, peu attractive. Dans un contexte sanitaire et sécuritaire dégradé, nous devons lutter contre la solitude du directeur d'école. Je pense aux drames survenus dans les écoles de Pantin et de Saint-Laurent-du-Var ; je pense également au mal-être de nombreux directeurs d'école, situés en première ligne pour honorer le service public d'éducation, malgré l'épidémie

soient aussi riches que les discussions en commission, avec cet esprit d'ouverture qui anime la Haute Assemblée. L'article 1 du texte prévoit d'accorder davantage de responsabilités au directeur d'école, en instaurant une délégation de compétences de l'autorité académique. permettrait un fonctionnement plus souple des écoles, sans pour autant revenir sur le lien hiérarchique avec le corps enseignant, qui relève de l'inspection de l'éducation nationale. L'article 2 fixe les conditions de nomination, d'exercice, d'avancement et de formation des directeurs d'école. il est proposé de renforcer les décharges de temps d'enseignement au profit des missions de direction. Une décharge totale est prévue pour les établissements à partir de huit classes, contre, actuellement, quatorze classes en élémentaire et treize en maternelle. En complément, les directeurs d'école seront libérés des trente-six heures consacrées chaque année aux activités pédagogiques complémentaires. J'appelle toutefois votre attention, monsieur le ministre, sur les risques de surcharge de travail pour les directeurs en cas de regroupement d'écoles. En matière de recrutement, la commission de la culture du Sénat a souhaité maintenir la possibilité de recourir à des enseignants volontaires ne figurant pas sur la liste d'aptitude, en cas de vacance du poste de directeur et en l'absence de candidature. Dans la mesure où une formation adaptée sera mise en place pour l'ensemble des directeurs d'école, nous sommes favorables à cette disposition visant à remédier de façon ponctuelle aux difficultés de recrutement. Toutefois, je voterai pour l'amendement de notre collègue Sonia de La Provôté tendant à faire en sorte que l'assistance administrative et matérielle ne relève que de l'État, et non des collectivités, car cela creuserait les inégalités entre les écoles, selon les moyens des communes. L'article 4 propose au directeur de contribuer à l'organisation du temps périscolaire, après avoir passé un accord avec la collectivité compétente. J'y suis favorable, dans la mesure où il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation, tant pour la commune que pour les directeurs d'école. Dans son ensemble, cette proposition de loi contribuera à l'amélioration des conditions de travail des directeurs d'école et à l'attractivité de cette fonction. Ces professionnels sont les premiers garants du bon fonctionnement des écoles et ils méritent cette reconnaissance spécifique. La parole

Ce texte n'est qu'une étape, mais c'est une étape attendue, que nous devons franchir, ce soir, au Sénat. Monsieur le ministre, nous saluons les mesures prises depuis 2017 : la mise en place d'un système d'accompagnement, le versement d'une prime de rentrée, l'amélioration des décharges dans les écoles de petite taille et le renforcement du rôle pivot du directeur dans le pilotage pédagogique. Une première réponse a été apportée aux besoins d'aides dans le cadre des parcours de préprofessionnalisation ; il faudra continuer d'avancer sur cette question essentielle. Notre commission a par ailleurs apporté un certain nombre de modifications. Elle a notamment voulu éviter l'émergence de tensions entre directeurs d'école et enseignants, en supprimant toute référence à l'absence d'une autorité hiérarchique des premiers sur les seconds.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je prends la parole au nom de Jacques Grosperrin, qui assiste cette après-midi, en compagnie du président Larcher, aux obsèques du sénateur honoraire du Doubs, Georges Gruillot, qui siégea sur nos bancs de 1988 à 2008.

insuffisamment compte, entre autres choses, des contrastes entre ville et campagne. Le directeur d'école ne figure ni dans la loi Guizot de 1833 ni dans la loi Falloux de 1850. Les termes d'« instituteurs » et d'« adjoints » sont en revanche présents dans la loi Duruy de 1867, signe de l'existence déjà établie de cette hiérarchie. L'article 10 de la loi Ferry de 1882 indique ce qui est dès lors la première raison d'être de la fonction : « Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence »,

on comptait plus de 47 000 directeurs d'école, dont 28 000 déchargés en partie de leur enseignement. Pour mémoire, les femmes représentaient alors 81,5 % des enseignants du premier degré et 73,2 % des directeurs.

un système de responsabilités sans reconnaissance ni moyens. Le directeur est un cadre intermédiaire indispensable, qui a su progressivement prendre sa place, mais qui n'a jamais été un chef d'établissement. Jusqu'à présent, sa fonction administrative se surajoutait à sa fonction d'enseignement, avec une formation quasi inexistante et considérée comme superflue. Le choix se portant sur des instituteurs et professeurs des écoles chargés d'une mission supplémentaire de direction, les inspecteurs choisissaient principalement des enseignants à la réussite pédagogique évidente, auxquels l'on ne proposait pas de formation spécifique ; était-ce une raison valable ? Il aura fallu attendre une note de service du 17 mars 1997 pour que soit véritablement souligné le besoin d'une formation au cours de la première année d'exercice. Tout cela a conduit, pendant trop longtemps, à une forme de solitude, souvent invoquée dans des conditions matérielles d'exécution difficiles. On surveillait les directeurs davantage que l'on ne les aidait, sans prendre en compte leur complexe polyvalence des tâches.

C'est l'organisation générale de notre enseignement primaire qui est en jeu au travers de ce texte, lequel doit répondre, en même temps, au mal-être trop souvent constaté de nos directrices et directeurs. Les objectifs du texte et de nos amendements sont donc clairs et volontaristes : renverser, positionner et conforter.

À ce titre, il nous semble inutile de créer une nouvelle instance, comme le conseil de la vie écolière ; les conseils d'école sauront s'adapter de façon souple. Il faut prévoir des conditions strictes et cohérentes d'accès à cette fonction, avec un avancement corrélé

Pour conclure, je souhaite rendre un hommage particulier à l'ensemble de la communauté éducative et aux directeurs d'école, qui ont su, pendant la pandémie, honorer leur mission. La parole

il me semble important de préciser que cette délégation ne concerne que le fonctionnement de l'école. Néanmoins, on ne comprend pas bien comment cette délégation sera déclenchée ni quels en seront les impacts concrets pour la communauté éducative. Cette solution permettra aux directeurs de disposer d'un pouvoir de fait sur les enseignants, dans le simple cadre de leurs fonctions au sein de l'établissement, pour assigner à ces derniers des missions nécessaires au bon fonctionnement de l'école, mais, en cas de refus d'un enseignant d'obéir au pouvoir délégué du directeur, désormais renforcé par la loi, que se passera-t-il ? Par ailleurs, le texte est muet sur la durée, la fréquence et l'amplitude de cette délégation : sera-t-elle permanente ? Sera-t-elle accordée au cas par cas ? S'appliquera-t-elle à toutes les questions de fonctionnement ? Sera-t-elle fondée sur un accord tacite ou sur des accords contractuels entre le directeur et l'autorité académique ?

que cette délégation de compétences ne sera pas automatique et de droit, et qu'il s'agira d'une simple possibilité. Notre amendement a donc pour objet de rendre la délégation de compétences de l'inspecteur d'académie vis-à-vis du directeur d'école dérogatoire, optionnelle et limitée dans son objet et dans sa durée.

Notre rapporteur nous a affirmé, lors de l'examen en commission, que cette précision serait de nature à jeter le doute, alors que la question des rapports entre directeurs et enseignants n'était pas abordée dans le texte. Or, à peine l'examen du texte en commission achevé,

Le directeur ne doit pas se placer au-dessus de l'équipe pédagogique ; il reste « un pair parmi ses pairs ». Les directeurs d'école sont d'ailleurs, dans leur quasi-totalité, très attachés à la notion de collectif et ont affirmé, à de nombreuses reprises, qu'ils ne souhaitaient pas un statut spécifique, question qui se profile derrière celle de l'autorité hiérarchique. Ce n'est pas en ouvrant une telle brèche que nous parviendrons à résoudre le sentiment de solitude et d'impuissance qui affecte souvent les directeurs d'école, ainsi que leurs difficultés à assumer l'ensemble de leurs missions. C'est pourquoi nous souhaitons que figure noir sur blanc dans la loi, la précision selon laquelle le directeur d'école, lui-même issu du corps enseignant, n'exerce aucune autorité sur les autres enseignants de son école, même dans le cadre de sa délégation fonctionnelle de compétences de l'inspecteur d'académie, comme cela a été voté très majoritairement à l'Assemblée nationale.

eh bien, écrivons-le clairement ! Cela permettra de délimiter le périmètre du cadre réglementaire qui s'appliquera à cette délégation de compétences. Cela permettra également à l'autorité académique de continuer de s'exercer sur la totalité des enseignants. Cela apaisera le débat, ce qui n'est pas forcément un luxe.

On voit bien les arguments que l'on peut donner dans un sens comme dans l'autre : j'entends ceux qui craignent les inconvénients d'une affirmation trop forte de la direction,

Cette autorité leur serait confiée dans le cadre limité de leur mission. Elle dépendrait non pas de leur personne, mais bien de la mission particulière qu'ils assument. Ainsi, elle serait limitée aux missions administratives et organisationnelles.

avec les représentants des organisations syndicales et avec le collectif des directeurs, car les lignes bougent. Tous constatent que le n'est plus tenable. Certains appellent même à la création d'un emploi fonctionnel de directeur d'école, et tous demandent une définition claire des missions que ce Cette disposition, qui modifie une organisation traditionnelle dont le besoin d'évolution fait pourtant consensus, fait écho à la réalité du fonctionnement quotidien d'une école. Un directeur d'école fait face, aujourd'hui, à des responsabilités croissantes, en particulier dans le champ de la sécurité. Il doit donc avoir les moyens de ses responsabilités et pouvoir les exercer en toute sérénité. Tel est le sens de cet amendement. Il n'y a aucune autre arrière-pensée ici que de permettre à un directeur d'école

le directeur ou la directrice, sur certains sujets, est en situation d'avoir une autorité pour jouer son rôle de responsable, au plein sens de ce mot, dans l'exercice de ses fonctions.

par trois références qui ne renvoient pas du tout à la situation que vous nous proposez. Ce que j'entends, moi, par « autorité fonctionnelle », c'est quelque chose qui pourrait emporter le rapport hiérarchique et le pouvoir de notation. On peut parfaitement considérer que, au titre de l'autorité fonctionnelle, le responsable d'établissement pourrait noter et avoir, de ce fait, un rapport hiérarchique sur les enseignants. D'où l'utilité de l'amendement précédent que vous avez rejeté. Si vous n'introduisez pas, dans l'autorité fonctionnelle, la nécessité du rapport hiérarchique, pourquoi nous avoir empêchés, tout à l'heure, d'indiquer clairement que cela ne faisait pas partie

On a basculé dans un système dans lequel vous instituez le chef d'établissement dans un rapport hiérarchique avec ses administrés que sont les membres de l'équipe enseignante. Il serait donc plus sage de revenir à la proposition de l'Assemblée nationale, parce que nous dérivons vers quelque chose qui n'a plus rien à voir.

J'ai connu, dans ma carrière d'enseignant, des directeurs qui étaient de véritables chefs d'équipe, de véritables lanceurs d'idées ou de projets. J'en ai connu d'autres qui auraient bien aimé être les directeurs que vous êtes en train de dépeindre aujourd'hui. Et je puis vous dire que c'est avec les

parce que j'ai l'impression que, dans ce débat, on ne veut pas dire les choses et que l'on tourne autour du pot. J'aimerais, cher Max Brisson, que vous nous disiez en quoi l'autorité fonctionnelle va apporter un plus à ce qui existe déjà

directrice d'école, que j'ai été confrontée, l'année dernière, à la mise en place du protocole de la crise sanitaire et que je rejoins parfaitement les propos de mon collègue Max Brisson

Mes chers collègues, j'entends que, dans les écoles, il y aurait des équipes d'enseignants formidables, où tout le monde s'entendrait et où la parole du directeur serait naturellement prise

que des instituteurs et des professeurs des écoles justifiant de trois années d'exercice dans des fonctions d'enseignement et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d'école. Cette disposition, à laquelle je souscris, emporte néanmoins des conséquences importantes pour l'enseignement privé sous contrat. Ainsi, il pourrait ne plus y avoir de direction unique pour une école primaire ou un collège. Un enseignant du second degré pourrait ne plus pouvoir diriger une école primaire privée sous contrat, ce qui existe dans les écoles privées sous contrat. Monsieur le ministre, je sais que ce sujet a été évoqué brièvement à l'Assemblée nationale et que vous aviez souligné qu'il relève du domaine réglementaire. Toutefois, sans assurance publique de votre part sur les conséquences de ces principes sur les directeurs d'école sous contrat, les craintes de l'enseignement privé continuent de grandir.

Cette question n'est pas anodine, puisqu'il est inscrit dans la loi que l'absence de fourniture de ces outils numériques créerait une situation d'illégalité. Une telle situation pourrait,, faire considérer au directeur qu'il n'est pas en capacité d'exercer ses fonctions, donc qu'il n'est plus tenu de le faire. Est-ce lui-même qui jugera du matériel nécessaire ? Est-ce la collectivité ? Est-ce sa hiérarchie ? Est-ce une circulaire ? Encore une fois, la réponse à cette question n'est pas anodine. Deuxièmement, la dotation en nouveaux outils numériques est susceptible de créer une charge supplémentaire. Ma question est simple charge doit-elle incomber ? Si les textes en vigueur sont suffisamment clairs concernant les réseaux informatiques, les biens immobiliers ou le matériel pédagogique, qui relèvent de la collectivité chargée de la compétence scolaire, il s'agit

Le texte issu de l'Assemblée nationale prévoyait que tous les directeurs bénéficieraient d'un avancement accéléré, aucune mesure de contingentement ne pouvant être opposée à leur avancement de grade. a justement supprimé cette disposition, qui risquait de créer une réelle embolie dans la promotion des professeurs des écoles, compte tenu du nombre de directeurs, le risque que seuls les directeurs puissent bénéficier d'avancement de grade. Cet amendement a pour objet de reprendre le dispositif voté par nos collègues députés en le réservant aux seuls directeurs des écoles de treize classes et plus, à savoir ceux qui bénéficient d'une décharge totale, soit 6 % de l'ensemble des directeurs. Il s'agit de prendre en compte la diversité des écoles et des directeurs et de trouver un juste équilibre entre revalorisation indiciaire des directeurs et mouvement de promotion des professeurs, qu'il ne faudrait

la faiblesse des dispositifs de formation se fait particulièrement sentir lorsqu'un directeur prend ses fonctions dans des écoles de grande taille, c'est-à-dire de plus de treize classes, fonctions auxquelles il consacre alors la totalité de son temps. cet amendement a pour objet d'instaurer une formation certifiante pour les directeurs des écoles de treize classes et plus. En revanche, la formation des autres directeurs ne revêtirait pas de dimension certifiante afin de ne pas réduire le nombre de professeurs pouvant postuler à cette fonction.

est à M. Max Brisson. Cet amendement vise à préciser l'objectif de la décharge pour les directeurs d'école. Si l'organisation effective des temps de décharge relève du décret, de nombreuses inquiétudes se sont

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, contre l'avis de votre rapporteur. Très